Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues,

Maire de Fréthun pendant vingt-deux ans, elle a mis toute son énergie et sa générosité au service de sa commune. Conseillère régionale des Hauts-de-France, cette cheffe d'entreprise fut une défenseure passionnée du Calaisis. Catherine Fournier s'est pleinement impliquée dans la vie démocratique de son département et de sa région, aux côtés de Xavier Bertrand. Cette femme de conviction devint sénatrice lors du renouvellement de 2017. Membre du groupe Union Centriste, elle est restée jusqu'au bout fidèle à son idéal humaniste et à son engagement au service des autres.

la commission des affaires européennes, puis la commission des affaires économiques, par sa connaissance des dossiers. Elle présida la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (Pacte) avec la plus grande rigueur.

Son sens politique, conjugué à son sérieux et à sa gentillesse, a marqué tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Elle s'est battue avec un courage incroyable contre la maladie, donnant en quelque sorte sens à l'espérance. Elle fut accompagnée avec tendresse et dévouement par son époux, sa famille et ses collègues. Je me souviens d'un échange récent que j'ai eu avec elle au téléphone elle me parlait des travaux de notre assemblée alors qu'elle partait une fois encore suivre le protocole de traitement. Au nom du Sénat tout entier- et bien au-delà -, -, j'exprime notre sympathie et notre profonde compassion à son époux, à ses enfants, à ses proches, au président et aux membres du groupe Union Centriste, ainsi qu'à tous ses collègues qui l'ont connu en commission. je vous propose d'observer un instant de recueillement.

Je vous remercie

la France s'active pour réhabiliter sur la scène internationale le prince saoudien assassin Mohammed Ben Salman ; pour vendre des Rafales à l'Égypte et aux Émirats arabes unis, qui serviront notamment à moderniser les bombardements de civils au Yémen. La France s'active pour participer aux préparatifs de la Coupe du monde en 2022 au Qatar, tout en fermant les yeux sur les 6 500 ouvriers esclaves morts sur les chantiers de ces stades pharaoniques à usage unique. La France s'active encore pour transmettre à l'Égypte des renseignements militaires, qui ont entraîné dix-neuf bombardements et la mort de milliers de civils. Quand l'alerte est lancée par un média indépendant, que fait la France ? Elle porte plainte pour violation du secret de la défense La France s'active pour honorer du plus haut grade de la Légion d'honneur le président al-Sissi pour l'ensemble de son oeuvre de piétinement des droits humains. Monsieur le Premier ministre, la France met aujourd'hui en oeuvre une cynique à l'efficacité douteuse, sur laquelle le Parlement est mal informé et peu consulté,

quoi qu'il en coûte

Je rappelle à la représentation nationale que notre politique d'exportation d'armes, sur laquelle portait votre question, est un pilier de notre diplomatie et de notre politique de défense

et international. Elle est conforme à nos engagements internationaux en matière de maîtrise des armements, de désarmement, de non-prolifération, de régulation du commerce des armes et d'interdictions relatives à certaines armes

Je pense aussi à la position commune 2008/944 de l'Union européenne définissant les règles régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires. Là encore, la France a été à l'initiative Dois-je vous rappeler également- surtout ici au Sénat ! -que le Gouvernement a porté la plus grande attention aux travaux conduits par Jacques Maire et Michèle Tabarot sur les exportations de matériels de guerre et de biens à double usage ? Nous avons adopté une série de mesures pour améliorer encore

apportée par le Gouvernement au Parlement. Il s'agit d'offrir une vision d'ensemble des priorités gouvernementales dans le domaine du contrôle des exportations des matériels de guerre et des biens à double usage. Dans ce cadre, cher président Gontard, nous revendiquons et nous assumons la signature récente d'un très important contrat prévoyant l'acquisition de 80 avions de combat Rafale par les Émirats arabes unis et de 12 hélicoptères

Je rappelle que ce contrat confortera plusieurs milliers d'emplois dans les 400 entreprises françaises oeuvrant pour le programme Rafale.

Et l'expression est faible ! À Esquelbecq, le niveau de l'eau a parfois atteint un mètre. Si ces secteurs doivent régulièrement affronter les conséquences de pluies abondantes, la récente pluviométrie, parfois cinquantennale, nous a rappelé qu'il convient d'être vigilant face à la puissance de l'eau ! Avant de poursuivre, je tiens à apporter mon soutien aux victimes de ces inondations, notamment à celles et ceux qui sont tétanisés à l'idée de réintégrer leur habitation, qui représente désormais un risque. Toutefois, je ne peux pas passer sous silence la remarquable mobilisation des services de l'État, des forces de l'ordre, des élus, des sapeurs-pompiers et des bénévoles pour secourir ces personnes dans un contexte d'extrême urgence.

Il est donc indispensable de procéder à un constat d'ensemble et de procéder à une analyse collégiale. Que penser du fonctionnement des wateringues, de l'état des matériels de pompage, d'un éventuel curage de l'Aa et des canaux non navigués et envasés ? Qu'en est-il des eaux situées en Belgique ? Quelle a été l'efficacité des bassins de rétention de crues ? Les façons culturales permettent-elles la percolation des terrains ? Les réponses seront multiples la solution résidera probablement dans un bouquet de propositions. Une chose est sûre : l'État devra faire un effort financier, car les collectivités ne peuvent plus tout supporter ! Madame la ministre, de nombreux maires déposent en ce moment leur dossier de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ils attendent une décision diligente.

vous l'avez rappelé, le département du Nord a connu un épisode pluvieux particulièrement intense les 27 et 28 novembre derniers, lequel a provoqué de nombreuses inondations et le débordement des rivières Yser et Lys,

qui feront l'objet d'un examen interministériel dès la semaine prochaine.

Avec la reprise des contaminations, la fréquentation de certains restaurants a chuté en seulement quelques jours. Pas moins de 50 % des repas et des fêtes de fin d'année sont d'ores et déjà annulés. Les discothèques sont contraintes de refermer leurs portes. C'est une véritable catastrophe pour ce secteur, qui entame sa période la plus importante de l'année et qui se remet à peine des conséquences des premières vagues du covid-19. Si les mesures de soutien du Gouvernement ont permis d'éviter le pire, ces entreprises ont vu leur trésorerie fondre comme neige au soleil.

Confirmez-vous une prise en charge à 100 % de l'activité partielle ? Allez-vous autoriser un nouveau report du remboursement des prêts garantis par l'État ? Comment comptez-vous compenser leurs pertes de chiffre d'affaires ? Vous avez annoncé hier une prise en charge intégrale des coûts fixes des entreprises, sans toutefois préciser le seuil de déclenchement de cette aide. Qu'en sera-t-il ? La

Monsieur le président, au nom du groupe Union Centriste, je vous remercie de l'hommage que vous venez de rendre à notre regrettée collègue Catherine Fournier. Ma question s'adresse à M. le ministre des outre-mer. Dimanche prochain, les Néo-Calédoniens sont appelés à se prononcer sur l'indépendance de leur territoire lors du troisième et dernier référendum d'autodétermination prévu par l'accord de Nouméa. Très vraisemblablement, pour la troisième fois, à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? », le « non » va l'emporter. l'emporter. Que se passera-t-il au lendemain du scrutin ? La question se pose avec d'autant plus d'acuité que les indépendantistes ont appelé à la non-participation et ont fait part de leur intention de ne pas reconnaître le résultat.

La société calédonienne est divisée. La Nouvelle-Calédonie doit retrouver une stabilité institutionnelle, seule à même de permettre de répondre à l'urgence économique et sociale et de régler les problèmes fondamentaux du territoire. Elle ne pourra pas y parvenir sans la France, qui devrait se saisir de ce moment historique pour enfin considérer ce territoire ultramarin à sa juste valeur.

Votre solution, qui consiste à proposer en priorité le vaccin Moderna, n'est pas de nature à rassurer celles et ceux qui sont réticents à se faire vacciner en raison des risques, certes très rares, inhérents à ce vaccin pour les moins de 30 ans. Aussi, ma question est simple : face aux ruptures de stocks de vaccins, où en est la production d'un vaccin français contre la covid-19 ? C'est honteux ! Le Gouvernement a investi 530 millions d'euros entre les mois de mars 2020 et de mars 2021 dans la recherche contre la pour quels résultats ? Certes, les dividendes des industriels du médicament ont progressé, mais où en sont les résultats de la recherche en France ?

Monsieur le ministre, nous l'avons déjà dit, il est urgent de lever les brevets et de réquisitionner Sanofi pour produire un vaccin public indépendant des intérêts des actionnaires. Face à cette crise sanitaire qui n'en finit pas, le Gouvernement est responsable de la situation des hôpitaux et du secteur médico-social, qui souffrent cruellement du manque de moyens humains et financiers. Au lendemain d'une journée de mobilisation nationale des personnels des structures associatives non lucratives, j'ai une pensée pour tous les oubliés du Ségur de la santé qui oeuvrent au quotidien qui oeuvrent au quotidien pour une société inclusive. Le renforcement de notre service public de la santé et du secteur médico-social doit constituer la priorité du prochain quinquennat.

question de l'assurance récolte est-elle plus que jamais d'actualité. Si l'épisode climatique du mois d'avril a montré qu'il était nécessaire de réfléchir à la diversification des exploitations ou de renforcer les dispositifs de protection, il a aussi mis en exergue le faible taux de souscription aux contrats d'assurance multirisque climatique.

d'un véritable enjeu de souveraineté. C'est pourquoi nous avons décidé, sur l'initiative du Président de la République et du Premier ministre, de proposer une réforme totale du système de couverture des risques. Songez, mesdames, messieurs les sénateurs, que, jusqu'à présent, nous avons laissé les agriculteurs se couvrir

un peu moins de 20 % de nos surfaces agricoles sont couvertes par un système d'assurance récolte, non pas parce que les agriculteurs sont des mauvais gestionnaires, mais parce que le système n'est pas suffisamment intéressant ni viable financièrement aux yeux des agriculteurs. Nous allons donc revoir tout le système.

un flot continu de propos fustigeant notre République, ses valeurs et ses principes, quinze jeunes, filles et garçons de notre pays,

a été souillée : des journalistes de l'émission Quotidien et de Mediapart ont été pris à partie, insultés, violentés et exfiltrés. La parole extrémiste, antirépublicaine, raciste et antisémite s'est libérée.

Monsieur le ministre de la santé, ma question fait suite à plusieurs interpellations et appels alarmistes de directeurs d'hôpitaux de ma région ces derniers jours. Une cinquième vague de la covid est en cours, dont on connaît déjà l'importance, mais pas encore la durée. Ce que l'on connaît bien en revanche, c'est ce que vivent nos hôpitaux depuis le début de la crise sanitaire. sont confrontés à la fois à une augmentation importante de leur activité, liée à l'épidémie, et à une baisse de leurs recettes du fait de la diminution ou du report des autres activités. À cela s'ajoute une crise majeure et structurelle de leur attractivité, à l'origine de difficultés de recrutement dans tous les services. Pour y répondre, du moins partiellement, le Gouvernement a mis en place la garantie de financement des établissements de santé, qui assure aux hôpitaux des recettes équivalentes à celles de l'année 2019. Or cette garantie expire à la fin du mois de décembre et nous n'avons aucune information sur son éventuelle prolongation. Au-delà de ce que représente une cinquième vague pour les hôpitaux, à savoir une pression accrue sur des personnels et des finances déjà exsangues, vous comprenez, monsieur le ministre, que cette incertitude pour l'année à venir accroît l'inquiétude des responsables hospitaliers. L'activité hors covid n'est jamais revenue à son niveau d'avant crise et, au vu des plans blancs qui se multiplient dans le pays, la situation ne va clairement pas s'améliorer. Aujourd'hui, pouvez-vous assurer aux établissements de santé qui nous en font la demande que vous prolongerez la garantie de financement, ce qui leur permettrait de souffler au moins jusqu'à la fin de cette cinquième vague

pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les centres de vaccination gérés par les maires ont parfaitement rempli leur rôle et ont permis de vacciner tous les Français qui le souhaitaient. L'annonce de la troisième dose a aussitôt entraîné une reprise de l'activité de ces centres. Or, à ce jour, beaucoup d'entre eux n'ont plus de créneaux disponibles avant la mi-janvier, et ce faute de vaccins et de personnels soignants en nombre suffisant. C'est le moment que vous avez choisi pour annoncer, sans aucune concertation avec les maires et en parfaite méconnaissance des impératifs logistiques auxquels ils sont confrontés, que les personnes âgées de plus de 65 ans pouvaient se rendre dans les centres de vaccination sans rendez-vous, et ce dès le lendemain de votre annonce. Bien sûr, je me réjouis de l'intérêt que les Français portent à cette troisième dose de vaccin, mais encore faut-il organiser

ils sont considérés comme la dernière roue du carrosse. Ce n'est pas correct ! Monsieur le Premier ministre, on a véritablement le sentiment que vous n'avez tiré aucun enseignement de vos erreurs : Paris décide toujours aussi seul On aurait pu penser que le Gouvernement allait enfin maîtriser ses annonces et engager une concertation avec les élus locaux et les personnels de santé qui mettent en oeuvre au quotidien la vaccination sur le terrain. Il n'en est manifestement rien.

pour eux, pas d'augmentation de 183 euros, pas de reconnaissance du travail accompli, contrairement à leurs collègues du secteur sanitaire et des En réaction à ces manquements, salariés et employeurs du secteur médico-social à but non lucratif, notamment du secteur du handicap, s'organisent. Partout en France, ils manifestaient le 30 novembre dernier. Ils scandaient leur colère face à un Ségur inachevé, à des inégalités de traitement injustifiées. Preuve de l'urgence et de la gravité de la situation, la mobilisation des employeurs est totale. En Dordogne, ils se sont rassemblés au sein d'un collectif pour défendre leurs salariés. Épuisés, découragés, désabusés, ces derniers fuient et se tournent vers des postes mieux rémunérés. Démissions, difficultés de recrutement, fermetures de places, de lits et, demain, d'unités entières : les craintes sont nombreuses. Monsieur le ministre, l'accompagnement et la sécurité des personnes en situation de handicap ne se résument pas aux soins. Or, aujourd'hui, leur prise en charge se dégrade. Le Ségur de la santé doit s'appliquer à l'ensemble des travailleurs du secteur social et médico-social. Combien de temps, monsieur le ministre, devront-ils encore attendre ? Combien de démissions, de postes vacants, de suppressions de services, d'interruptions ou de refus d'accueil vous faudra-t-il pour réagir ?

La veille de cet hommage, le 14 octobre, Jean-Christophe Peton, professeur dans le Jura, a osé s'exprimer, en réponse à un message laconique de son proviseur sur l'application Pronote annonçant la minute de silence en hommage

Je suis désolée, monsieur le ministre, mais vous ne m'avez vraiment pas convaincue ! Alors que ce sont la peur, la lâcheté et le manque de courage qui ont conduit à la mort de Samuel Paty, ce professeur qui défendait la liberté d'expression, force est de constater que, dans votre ministère, on continue à ne pas nommer les choses. En un an, monsieur le ministre, rien n'a changé. Dans quelques semaines, comme vos collègues, vous devrez présenter votre bilan aux Français. Or, malheureusement, cette merveilleuse institution qu'est l'éducation nationale n'aura jamais autant été remise en cause depuis cinq ans,

des agences et des éditeurs de presse, sous peine de se voir appliquer des astreintes pouvant aller jusqu'à 900 000 euros par jour de retard. Cette double décision sanctionne clairement la société Google, qui n'avait eu de cesse, depuis le vote de la loi du 24 juillet 2019, de tenter de la contourner pour ne pas payer ces droits Cette double décision a été unanimement saluée par les acteurs du secteur, en raison de sa fermeté et de son caractère exemplaire.

a-t-elle payé l'amende de 500 millions d'euros ? Lui a-t-on appliqué les pénalités d'astreinte, alors que la période de négociation est désormais achevée depuis un peu plus d'un mois ?

Par ailleurs, l'Autorité de la concurrence a ordonné à Google de se conformer à deux injonctions prononcées dans sa décision initiale, sous peine d'astreintes journalières. La société Google a donc été sommée d'entrer en négociation de bonne foi avec les éditeurs et les agences de presse qui le désirent et de communiquer les informations nécessaires

La balle est aujourd'hui dans le camp des éditeurs. C'est à eux de décider s'ils souhaitent continuer de négocier ou s'ils

(PLU) des communes rurales se trouvent ainsi amputés de 60 % de surfaces constructibles. Les citoyens désireux de construire sont mécontents ; les maires excédés par une administration raide et tatillonne.

Projet d'extension d'un bâtiment agricole pour valoriser une activité économique de bois : refus ! À l'heure où la crise sanitaire entraîne un retour à la campagne des citadins, nos villages ne veulent pas être condamnés. Ils ne veulent pas être les faire-valoir et les boucs émissaires d'un urbanisme débridé. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, quelles solutions allez-vous mettre en oeuvre afin de ne plus condamner injustement nos villages ?

L'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal ou, mieux, d'une carte communale- un document très simple -permet de s'affranchir du règlement national d'urbanisme et de retrouver des capacités à construire.

ils veulent de la souplesse dans l'application de la loi Montagne ; ils veulent un équilibre intelligent et pragmatique entre l'objectif de zéro artificialisation nette et un urbanisme sauvage.

en tant qu'industrie hyper électro-intensive des coûts de fourniture d'énergie plus élevés que ses principaux concurrents européens ou chinois. D'autre part, elle a dû faire face au cours des dernières années à la concurrence déloyale de la Chine, qui a entraîné une baisse de ses prix, alors même que les autres États se sont protégés de façon efficace, grâce à des mesures antidumping beaucoup plus fortes qu'en Europe. À titre d'exemple, les droits antidumping sont de 17 % en Europe, contre 53 % en Australie et 122 % aux États-Unis.

emploi et savoir-faire

et trouver des solutions pour l'ensemble de ses sites industriels français. Comme vous le savez, Ferropem a subi une restructuration financière particulièrement importante, à l'échelle mondiale, laquelle a pesé sur le devenir de ses sites.

Jean-Charles Colas-Roy, Anthony Cellier, Vincent Rolland, Hervé Gaymard, Émilie Bonnivard, Marie-Noëlle Battistel, et j'en oublie certainement

sénatrice, nous allons continuer à accompagner cette industrie, qui, vous avez raison de le souligner,

Certains centres hospitaliers, dont celui de Cherbourg, dans la Manche, ont dû réactiver le plan blanc et ont déprogrammé les interventions médicales non urgentes. La fragilité structurelle de ces établissements hospitaliers préexistait avant cette nouvelle vague épidémique. En effet, dans certains territoires, être admis aux urgences est devenu un parcours du combattant ! Au cours des derniers mois, de nombreux services ont été poussés à la fermeture, faute de personnel soignant et de médecins.

La direction a dû faire appel à des intérimaires, ce qui ne permet pas un fonctionnement optimal du service, au grand désarroi des médecins titulaires. Certes, le Ségur de la santé était nécessaire, mais il montre déjà ses limites puisque les personnels manquent, quittent le service public ou refusent d'y travailler. Vous nous avez annoncé des financements exceptionnels en matière d'investissements. Or c'est le fonctionnement ou l'attractivité de l'hôpital public qui est en cause. Si le rôle de l'État est de protéger la population contre la covid-19, celui-ci doit également assurer une couverture sanitaire homogène et équitable, notamment dans les territoires ruraux. ruraux. Malades, sachez-le : vous n'avez pas la même chance d'être soignés selon que vous habitez dans une ville littorale au sud de la France ou dans une petite commune rurale, aussi charmante soit-elle

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le ministre, je connais votre attachement au principe de l'école inclusive et je salue le fait que vous ayez élevé au rang de priorité un meilleur accompagnement à l'école des enfants en situation de handicap. politique est partagée par tous les maires, notamment par ceux des plus petites communes. Toutefois, l'arrêt du Conseil d'État du 20 novembre 2020 vient fragiliser une telle politique. En effet,

Se pose aussi la question de leur capacité à supporter cette nouvelle charge, notamment sur le plan financier., cette évolution pourrait remettre en cause l'équité territoriale en matière d'accueil des enfants handicapés, qui ne peut dépendre de la seule capacité financière des communes. Une école réellement inclusive ne peut pas et ne doit pas faire l'impasse sur la continuité des temps scolaires et périscolaires.

Enfin, peut-on envisager de prendre le temps de clarifier les financements permettant un accompagnement pérenne des élèves en situation de handicap, afin que ceux-ci ne dépendent pas uniquement des communes ? La parole

rupture sur le terrain, y compris au mois de janvier prochain. Aucun enfant ne doit se trouver dans une situation désavantageuse du fait de cette nouvelle définition juridique. Nous en

pour examiner la proposition de loi visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer, je souhaite

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, M. le ministre de l'intérieur m'a fait connaître que, en application de l'article L.O. 320 du code électoral, Mme Amel Gacquerre est appelée à remplacer, en qualité de sénatrice du Pas-de-Calais, Catherine Fournier, décédée le 7 décembre 2021. Son mandat a débuté le mercredi 8 décembre 2021, à zéro heure. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 27 voix pour, 2 voix contre la nomination de Mme Anne-Claire Mialot en tant que directrice générale de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle est parvenue à l'adoption d'un texte commun.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

ce sujet qui m'est cher, comme vous le savez peut-être, et auquel personne ne peut rester indifférent. Nous avons eu l'occasion de débattre régulièrement, dans cet hémicycle comme à l'Assemblée nationale, nationale, d'une meilleure prise en charge des enfants malades et de l'accompagnement de leurs familles. Nous avons ainsi abordé le financement de la recherche sur les cancers pédiatriques et débattu d'un texte, que j'ai défendu en tant que députée, visant à renforcer la prise en charge de ce type de cancers par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels ou encore le droit à l'oubli. Nous avons été plusieurs à porter au débat national les sujets si nécessaires à l'accompagnement des familles en situation de fragilité.

pour permettre, notamment, le doublement de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). Ces textes ont permis de véritables avancées et amélioré l'accompagnement des malades et de leurs proches. Je souhaite bien sûr saluer le travail remarquable et l'engagement de Béatrice Descamps et de Jocelyne Guidez, qui ont toutes deux porté le travail parlementaire sur ces textes dans leur assemblée La proposition de loi visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer tend à ouvrir des jours de congé aux parents et à faciliter le parcours de santé et la scolarité des enfants malades. Sur ce sujet si douloureux, l'éducation nationale n'est pas en reste. Elle prend toute sa part pour accueillir ces élèves et les quelque 11 000 d'entre eux qui sont scolarisés dans des établissements hospitaliers ou sanitaires. des dispositions sont prévues pour permettre aux enfants et aux adolescents dont l'état de santé rend nécessaire l'administration de traitements médicaux particuliers de poursuivre une scolarité dans les meilleures conditions possible. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation légale, prévue dans le code de l'éducation.

Les modalités en matière d'examens et de concours des candidats sont définies dans une circulaire de décembre 2020, qui assure une cohérence entre les aménagements de scolarité inscrits dans le PAI et les demandes d'aménagement des épreuves d'examen. Enfin, nous ne pouvons aborder cette proposition de loi sans évoquer les remarquables progrès enregistrés au cours des dernières années en matière de scolarisation des enfants porteurs d'un handicap, pour une école plus inclusive. Je veux saluer, à cet égard, la politique volontariste de Jean-Michel Blanquer et de ma collègue Sophie Cluzel. Dans certains cas, les enfants malades ne peuvent pas se rendre en milieu scolaire, parce qu'ils sont hospitalisés ou contraints de rester à leur domicile. existe alors plusieurs solutions. Parfois, c'est l'école qui vient à eux. Ainsi, près de 800 enseignants spécialisés sont affectés dans les hôpitaux ou dans des maisons d'enfants à caractère sanitaire.

au milieu d'un magnifique parc, une très belle école, colorée comme toutes nos écoles, à la différence près que les élèves arrivent le matin en classe en fauteuil roulant ou avec une perfusion au bras. Je profite de cette intervention pour les saluer, mais aussi pour saluer et remercier leurs professeurs. Lorsque les élèves doivent rester à leur domicile, ce sont les enseignants qui viennent à eux afin de leur permettre de conserver un lien avec leur école et leur classe.

Ce programme est destiné aux élèves empêchés par une maladie grave ou de longue durée et désireux de suivre des cours à distance à l'hôpital, en établissement de soins ou à domicile, voire sur leur lieu de convalescence. Il est destiné à améliorer l'accompagnement pédagogique et la socialisation des jeunes élèves ou des étudiants éloignés de leur classe. Il prend des formes diverses, depuis une petite caméra posée sur le bureau du professeur, jusqu'à un robot, de la taille d'un enfant, placé au milieu de la classe. Vous l'aurez compris, le ministère de l'éducation nationale prend toute sa part et répond aux besoins des élèves présentant des particularités de santé ou des maladies graves, comme le cancer. C'est notre responsabilité, bien sûr, et ce qui fait la grandeur de l'école de la République. Au-delà des normes juridiques, textes, règlements, outils, mesures, dispositifs, nous avons, avant tout, une obligation morale. morale. Épreuve intime et douloureuse qui bouleverse des familles et des fratries, la maladie, particulièrement le cancer, suscite un sentiment d'injustice, qui se transforme souvent en révolte lorsqu'elle touche nos enfants. Nous ne saurions être indifférents à la charge psychologique des parents concernés, qui deviennent des aidants familiaux, ni à la fragilité et aux difficultés des enfants. des enfants. Je l'évoquais dans mon propos introductif, à travers ces textes successifs- s'il fallait en apporter la preuve, je crois que c'est fait -, nous sommes tous plus que jamais mobilisés pour lutter contre les inégalités, pour soutenir les plus fragiles, nos enfants malades et leur famille. C'est aussi ce qui fait l'honneur et la grandeur de notre société. J'aime beaucoup cette citation de Pythagore : « Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant ».

je tiens tout d'abord à m'associer à l'hommage qui a été rendu par le président Larcher à notre collègue Catherine Fournier, qui nous a quittés hier. La proposition de loi que nous examinons vise à faciliter la scolarisation et l'accompagnement par leur famille des enfants atteints d'une pathologie chronique ou d'un cancer. Déposée par notre collègue députée Béatrice Descamps, elle a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en première lecture le 25 mars dernier. Son premier objectif

Le droit existant permet déjà aux salariés et aux agents publics de s'absenter de leur travail pour faire face à diverses situations liées à la maladie ou au handicap d'un enfant. et à la sécurisation des parcours professionnels, d'un congé d'au moins deux jours à l'annonce de la survenue d'un handicap chez leur enfant. Il est rémunéré par l'employeur et assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des congés annuels. Par ailleurs, lorsque l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, les salariés bénéficient, d'une part, du mécanisme de don de jours de repos un parent d'un enfant gravement malade et, d'autre part, d'un congé de présence parentale. Rappelons également que, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite une hospitalisation immédiate après sa naissance, la première période de quatre jours de congé de paternité et d'accueil est prolongée de droit dans la limite de trente-deux jours consécutifs. Enfin, le salarié bénéficie de trois jours par an en cas de maladie ou d'accident de l'enfant à charge de moins de seize ans. Cela permet à un parent salarié de s'absenter en cas d'annonce de la maladie de son enfant, mais l'employeur n'est pas tenu de le rémunérer. Les agents publics bénéficient quant à eux d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à certains événements familiaux. Par ailleurs, le congé de présence parentale est également prévu pour les fonctionnaires et le don de jours de repos leur a été étendu par décret. La survenance d'une maladie chez l'enfant est un choc brutal et imprévisible, qui nécessite une réaction immédiate de sa famille. Pour les parents, qui ont besoin d'un temps pour s'organiser et appréhender la pathologie, le travail constitue le premier obstacle : si la majorité des employeurs se montrent compréhensifs, il existe des inégalités qui justifient la création d'un congé spécifique. L'article 1 de la proposition de loi crée donc un nouveau motif d'absence pour événement familial au bénéfice des salariés en étendant le congé de deux jours accordé pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant aux cas de pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer. Il inscrit par ailleurs dans la loi le principe d'une autorisation spéciale d'absence pour les fonctionnaires dans les mêmes cas. Le décret qui précisera la liste des pathologies chroniques concernées devra être pris rapidement- j'insiste sur ce point. Comme les autres congés pour événement familial, celui-ci serait à la charge de l'employeur. Ce dispositif, qui constitue l'apport le plus substantiel de la proposition de loi, permet de combler une lacune des différents congés existants. La commission vous propose donc de l'approuver. Le deuxième objectif de ce texte est de développer des échanges entre les parents et l'équipe éducative afin d'améliorer les conditions de travail de l'enfant à l'école. Conformément au principe de scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction, les enfants, adolescents et adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant peuvent être scolarisés au sein de dispositifs adaptés. En particulier, un projet d'accueil individualisé peut peut être mis en place lorsque la scolarité de l'élève nécessite des aménagements. Ce document précise la nature de ces aménagements, notamment la conduite à adopter en cas d'urgence. Les principales pathologies concernées sont l'asthme, les allergies, le diabète et l'épilepsie. Les cancers, leucémies et tumeurs, plus rares, représentent une bien moins grande proportion des PAI. Ces aménagements sont élaborés avec le concours du médecin scolaire ou de la protection maternelle et infantile, à la demande de la famille ou, en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Les échanges entre parents, enseignants, médecins scolaires, nécessaires à cette élaboration, ont été récemment renforcés par la circulaire du 10 février 2021, laquelle prévoit notamment des réunions d'information censées impliquer l'ensemble des parties prenantes. Elles peuvent pourtant parfois être insuffisamment inclusives et se tenir dans un délai trop long, entraînant retard et incompréhension chez certains professionnels, qui peuvent, en fin de compte, refuser de signer le PAI. Pour répondre à ces difficultés, l'article 2 prévoit l'organisation d'une réunion portant sur les modalités de mise en oeuvre du PAI. Celle-ci devra rassembler l'élève, ses responsables légaux, le directeur ou le chef d'établissement, ainsi que l'enseignant ou le professeur principal. Pourront y prendre part d'autres professionnels accompagnant l'enfant sur le temps scolaire ou périscolaire, un représentant de la collectivité territoriale compétente, ainsi qu'un professionnel de santé ou de la médecine scolaire. Elle devra se tenir si possible dans un délai de vingt et un jours à compter de l'annonce du diagnostic ou en amont de l'arrivée de l'enfant dans l'établissement. L'article 2 améliore en outre l'information des enseignants grâce à une documentation. Le retour à l'école peut être difficile pour l'enfant, surtout lorsque son aspect physique est modifié par la maladie. Les progrès considérables déjà observés, grâce notamment aux robots de téléprésence, seraient utilement complétés par le temps d'échange prévu à l'article 2, mené mené conjointement par un intervenant du secteur médical ou associatif et le professeur et organisé à la demande des parents. L'enjeu est de préparer la classe au retour de l'enfant à la suite d'une hospitalisation ou d'une absence prolongée à cause d'une pathologie chronique ou d'un cancer. Au-delà de ces dispositions, j'attire l'attention du Gouvernement sur l'amélioration de l'équipement des établissements du premier degré en stylos auto-injecteurs. Ces dispositifs, déjà imposés dans les établissements du second degré, sont très utiles en cas de réaction anaphylactique et peuvent empêcher la survenance

constituent un axe d'amélioration certain. L'article 2 prévoit donc d'étendre aux maladies chroniques la formation spécifique des enseignants de l'éducation physique et sportive sur les différentes formes de handicap,

Ces dispositions s'appuient sur les outils existants pour combler les lacunes de la formation du personnel enseignant et d'éducation. En pratique, il serait pertinent d'ouvrir aux enseignants chargés d'enfants malades certains modules de formation, très complets, destinés aux enseignants spécialisés dans le cadre du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive. En ce qui concerne les conditions de passation des examens, sujet important, des aménagements particuliers sont déjà prévus pour les élèves en situation de handicap ou atteints de troubles de la santé invalidants. Ces contextes de fort stress sont propices aux crises, face face auxquelles il faut savoir réagir. Pourtant, les centres d'examen ne sont pas toujours informés de la présence d'élèves bénéficiant d'un PAI ni du contenu de celui-ci. L'article 3 prévoit donc la communication du PAI au centre d'examen lorsque celui-ci est distinct de l'établissement d'origine de l'élève. Il peut y être indiqué si la présence d'un professionnel de santé est nécessaire. Mes chers collègues, comme l'a relevé la commission, cette proposition de loi soulève d'importantes questions, auxquelles elle n'apporte que des réponses modestes. Ses dispositions concernant l'école n'ont, en réalité, pas besoin d'un texte législatif pour être mises en oeuvre, et l'on peut se demander, madame la secrétaire d'État, ce qui empêche le Gouvernement de s'y employer, alors qu'il soutient cette proposition de loi. Celle-ci s'ajoute à une série d'autres textes ponctuels portant sur des sujets connexes sur lesquels une vision globale semble encore faire défaut. Ce texte représente néanmoins une avancée et répond à une certaine urgence pour les associations de parents. Son adoption conforme permettra l'entrée en vigueur rapide de l'article 1 et facilitera, en définitive, la vie des familles concernées par la maladie chronique d'un enfant. La commission vous propose donc de l'adopter sans modification. La parole

Une telle disposition existe déjà pour l'annonce de la survenue d'un handicap depuis l'adoption de la loi du 8 août 2016. L'extension de ce congé exceptionnel à l'annonce d'une maladie chronique telle que le diabète ou d'un cancer permettra de laisser quelques jours à la famille pour s'organiser et effectuer l'apprentissage thérapeutique nécessaire à la compréhension de la maladie. Cette annonce est souvent brutale et nécessite un temps d'adaptation et d'échange spécifique avec l'enfant et les professionnels. Ce congé serait rémunéré par l'employeur et les maladies concernées seraient précisées par décret. La proposition de loi prévoit également d'améliorer l'accompagnement de l'enfant dans sa scolarité après l'annonce de sa maladie. Ce sont des dispositions de nature réglementaire, mais nous comprenons parfaitement la volonté de l'auteure

Ce dispositif prendra la forme d'une réunion entre l'élève, les parents et l'équipe pédagogique dans les vingt et un jours à compter de l'annonce du diagnostic. Il me paraît particulièrement important, compte tenu du manque de formation et d'information des enseignants sur la prise en charge d'enfants atteints de maladies graves ou de certaines pathologies chroniques méconnues, telles que l'épilepsie. Si le quotidien des familles est bouleversé par l'annonce de la maladie, les enseignants sont souvent désemparés, notamment les professeurs d'éducation physique et sportive. La prise en charge de l'enfant doit être anticipée, organisée et adaptée, tout comme l'accompagnement des enseignants. Ces enfants doivent faire l'objet d'une attention particulière, en raison de leur maladie, mais également pour prévenir toute situation de harcèlement ou de mise à l'écart à la suite d'une crise. L'article 3 prévoit l'information systématique du centre d'examen de la présence d'élèves disposant d'un projet d'accueil individualisé afin qu'il puisse prendre ses dispositions en amont de leur accueil et prévoir, par exemple, la présence d'un professionnel de santé. Ces dernières années, de nombreuses mesures ont contribué à renforcer l'accompagnement des enfants atteints de maladies graves. Le Sénat a ainsi adopté récemment la proposition de loi de Paul Christophe, député du Nord, visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu. Je pense également à la proposition de loi de mon collègue nordiste Guy Bricout. Au même moment, le Gouvernement a revalorisé à hauteur du SMIC le montant de l'allocation journalière versée dans cette situation. Ces démarches participent, d'un même tenant, à rendre notre société plus juste et plus solidaire. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires votera cette proposition de loi.

réunis dans cet hémicycle pour examiner la proposition de loi visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer, je souhaite tout d'abord remercier Mme la députée Béatrice Descamps, avec qui j'ai pu échanger, pour le travail accompli et le volontarisme qu'elle a su insuffler dans nos deux chambres sur ce sujet. Accompagner ces familles est un devoir ; il est impossible d'en refuser la responsabilité en notre qualité d'élu. Nous devons les aider en leur donnant les moyens de continuer à vivre aussi normalement que possible dans une telle situation. Si l'école n'est pas aussi inclusive que nous pourrions le souhaiter, des efforts significatifs, même s'ils sont encore loin d'être suffisants, ont été faits pour les enfants présentant un handicap. fait- ou trop peu -pour les enfants porteurs d'une maladie chronique ou d'un cancer. Les enseignants ont besoin de connaître et de comprendre les conséquences, les répercussions de la maladie ou du traitement sur la scolarité de l'élève, sur sa capacité d'attention, de concentration, sur sa fatigabilité, et ce afin d'adapter au mieux leur pédagogie. L'introduction d'un congé spécifique, à l'instar de celui dont bénéficient les parents d'enfants atteints d'un handicap, est une avancée indéniable, un progrès dont nous ne pouvons que nous féliciter. Toutefois, les échanges et les rencontres sur le terrain nous ont permis de mesurer les attentes de nos concitoyens touchés par cette tragédie. Ce que nous devons retenir est simple : bien évidemment, deux jours, ce n'est pas assez, et, bien sûr, il faudra faire plus et encore mieux pour ces enfants et leurs parents. Deux jours, c'est court. Deux jours, c'est peu pour encaisser le choc. L'annonce d'un tel diagnostic est toujours un moment difficile et douloureux pour les familles. Si certaines pathologies ne nécessitent pas d'hospitalisation ou d'apprentissage thérapeutique particulier, d'autres requièrent en revanche une hospitalisation immédiate. Les parents et les enfants doivent alors comprendre la maladie et apprendre à la gérer, à repérer certains signes, à administrer des traitements, à utiliser du matériel médical, par exemple à faire une injection ou à utiliser un lecteur de glycémie. L'enfant a besoin de la présence de ses parents pour le suivi de la maladie, mais aussi pour le rassurer. Je profite de cette intervention pour saluer le travail titanesque effectué par nos associations. À titre d'exemple, je citerai la Ligue contre le cancer, qui, au-delà de toutes ses actions, accompagne et soutient les parents d'enfants malades. Dans mon département des Alpes-Maritimes, l'association Adrien, dont je suis la marraine, oeuvre au quotidien pour soulager les familles se bat avec de modestes moyens pour récolter des fonds et mener des projets. Au printemps prochain, la maison d'Adrien verra le jour, un lieu unique en France destiné notamment à héberger les familles dont l'enfant est hospitalisé. Il y a là aussi un sujet.

Cette reconnaissance législative des enfants atteints d'une maladie chronique et de leurs parents constitue une première pierre. Pour conclure, je m'adresserai à Adrien, Flavien ou Paloma nous ne cesserons jamais de travailler pour aller plus loin et répondre avec justesse aux cris d'alarme des familles, qui affrontent avec courage la maladie de leur enfant et les peurs qui en découlent inévitablement. inévitablement. Fidèle à mon engagement de toujours, je suis fière d'appartenir à une majorité qui s'investit dans la protection et la défense des familles frappées par la maladie. C'est donc en cohérence que je soutiens la création d'un congé spécifique, qui est nécessaire tant du point de vue du droit que du point de vue humain.

L'établissement d'un lien étroit entre santé et environnement est ancien. Hippocrate écrivait dans son traité « Pour approfondir la médecine, il faut d'abord considérer les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. » Les écologistes font d'ailleurs ce constat depuis toujours. En 2007, dans son ouvrage, le toxicologue André Cicolella a marqué les esprits en parlant de « pandémie des maladies chroniques

cet égard, je ne peux que rappeler l'importance de développer des recherches multidisciplinaires sur les maladies chroniques sous un angle médical, mais aussi social, économique et environnemental. santé définit la maladie chronique comme un « problème de santé qui nécessite une prise en charge sur une période de plusieurs années [ ...], engendrant un besoin de soins médicaux, d'aide psychologique, d'éducation ou d'adaptation Aussi cette proposition de loi vise-t-elle à mieux accompagner les enfants atteints de ces pathologies en milieu scolaire, ainsi que leur entourage. Elle est bienvenue sur un aspect notable : le congé de deux jours qu'il est prévu d'inscrire dans le code du travail pour les parents qui apprennent que leur enfant est atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer. Deux jours, cela peut sembler modeste ; néanmoins, la reconnaissance de ce droit nouveau marque une réelle avancée, qu'il conviendra d'étendre, y compris par les accords de branche. nous nous interrogeons sur l'ambition de l'article 3, raboté par rapport à sa version initiale. Ainsi, la présence « obligatoire » d'un médecin ou d'un infirmier scolaire dans chaque centre d'examen durant les épreuves, d'assurer l'équité des conditions de travail entre les élèves, devient une présence « souhaitable » dans la rédaction qui nous est proposée. De fait,

L'éducation et l'apprentissage thérapeutiques nécessitent que soient déployés au sein de l'éducation nationale des moyens humains à la hauteur. Le Gouvernement a récemment demandé au député Paul Christophe de formuler dans un rapport des propositions d'amélioration des dispositifs existants.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je remercie à mon tour le groupe Union Centriste d'avoir déposé cette proposition de loi, qui concerne entre 1,5 million et 4 millions d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes âgés de quelques

Il viendrait également en complément de la proposition de loi que nous avons votée le 4 novembre dernier visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu. Sur le fond, cette proposition de loi vise tout d'abord à mieux accompagner les enfants malades dans le milieu scolaire. Nous savons combien c'est important. La crise sanitaire n'a fait que conforter ce constat. Ainsi, il s'agit de maintenir la continuité pédagogique des apprentissages scolaires pour des enfants soumis à des interruptions de scolarité lors des examens médicaux et en raison des effets secondaires de leur maladie et de ses traitements. Il s'agit également de lutter contre les préjugés et les stéréotypes que subissent ces enfants malades. Il s'agit enfin de veiller à l'aménagement des épreuves des examens de ces enfants. Initialement, la proposition de loi prévoyait la présence d'un médecin ou d'une infirmière scolaire dans le centre d'examen, mais, face au manque de personnels, l'Assemblée nationale a préféré faciliter la communication du projet d'accueil individualisé.

Nous regrettons également que les services d'éducation spéciale et de soins à domicile ou encore les aidants familiaux- c'est là la limite de cette proposition de loi -ne soient pas mobilisés dans les dispositifs existants.

Selon une enquête réalisée en 2016- en 2021, les chiffres devraient être plus accablants -, le reste à charge moyen annuel pour un malade chronique s'élève à 752 euros.

je tiens à saluer la députée Béatrice Descamps, présente dans nos tribunes, pour son travail auprès des familles dont les enfants sont porteurs de maladies graves, ainsi que pour son engagement en faveur d'une meilleure prise en charge de la scolarisation de nos enfants. Le groupe Union Centriste aura eu raison d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de nos travaux. Je remercie aussi notre collègue et rapporteur Alain Duffourg pour la clarté de son rapport. Apprendre que son enfant est porteur d'une maladie grave ou handicapante représente évidemment pour les familles une préoccupation certaine, voire un choc psychologique selon les cas. Ces familles apprécieront de savoir que le Parlement oeuvre afin qu'elles puissent bénéficier de deux jours de congé lorsqu'elles apprennent que leur enfant est atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer. La durée de ce congé, qui pourrait être perçue comme symbolique, est avant tout une avancée. Le travail est l'un des premiers obstacles qui empêchent les familles de prendre du temps pour se remettre de leurs émotions, mais aussi, et surtout, pour s'organiser, se renseigner, effectuer les démarches nécessaires, être conseillées et accompagnées.

en étendant le droit à congé jusqu'ici réservé aux parents apprenant le handicap de leur enfant aux parents apprenant la pathologie chronique ou le cancer de leur enfant.

Nous serons très attentifs à ce qu'aucune pathologie ou maladie grave ne soit oubliée. Oublier une seule des pathologies chroniques, c'est négliger certaines familles, c'est négliger l'enfant porteur de la maladie. Puisque j'évoque le décret, madame la secrétaire d'État, pouvez-vous prendre l'engagement

des mêmes chances de réussite. La maladie ne doit pas être un frein à la scolarité et à l'épanouissement des enfants. L'article 2 prévoit un échange entre l'ensemble des personnes impliquées afin d'évoquer les conséquences possibles de la maladie ou des traitements,

Proposer aux intervenants de la documentation thématique afin de leur permettre de mieux appréhender les conséquences de la maladie sur la scolarité va dans le bon sens. Adapter les dispositifs d'aménagement des classes, mettre en oeuvre des formations de sensibilisation à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, engager la formation spécifique des enseignants d'éducation physique et sportive sur les différentes formes de handicap, c'est rendre l'école plus inclusive. En ce qui concerne l'école, nous regrettons vivement que l'article 44 alinéa 3 et l'article 45 de la Constitution ne puissent permettre, dans le cadre de cette proposition de loi, une réflexion sur la médecine scolaire.

et environ 2 500 enfants sont atteints d'un cancer. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui aborde un sujet douloureux, qui ne peut laisser personne indifférent. La maladie

Un enfant malade a plus que quiconque besoin d'une vie sociale riche et équilibrée. Je tiens à saluer le dispositif mis en place à l'article 1, qui l'article 1, qui vise à répondre à la difficulté, pour les parents, de concilier vie privée et vie professionnelle lorsque survient la maladie de leur enfant. En effet, une telle annonce est toujours une épreuve difficile à surmonter pour les familles. Ce nouveau droit ne règle évidemment pas tout deux jours peuvent sembler dérisoires pour certains, mais c'est toutefois une avancée. Le groupe du RDSE soutient évidemment cette disposition, car il faut laisser du temps aux parents pour commencer à accepter cette annonce et, surtout, pour mieux s'organiser dans leur quotidien. Ce texte entend également améliorer l'accueil de ces enfants à l'école. Si la scolarisation des enfants en situation de handicap a progressé ces dernières années- le taux de scolarisation a été multiplié par trois depuis la loi de 2005 -, celle des enfants porteurs de maladies chroniques reste encore trop faible. C'est pourquoi la formation des équipes pédagogiques aux pathologies chroniques est une très bonne chose. Trop d'enseignants, souvent par crainte de mal faire, sont en effet réticents à accueillir ces enfants. Les former et les sensibiliser permettra à ces enfants de bénéficier d'une scolarité normale et d'un accompagnement mieux adapté à leur état de santé. Je me félicite tout particulièrement de l'article 2 , qui permettra de faciliter la réintégration de l'enfant malade en milieu scolaire. Le retour à l'école reste en effet un moment particulièrement difficile lorsque l'enfant est frappé par la maladie. Permettre un réel temps d'échange au sein de l'établissement avec les élèves de la classe pour leur expliquer la situation, avant le retour de leur camarade, devrait permettre de retisser le lien social autour de l'enfant malade, ce qui lui donnera l'énergie indispensable pour se battre contre la maladie. Bien que nous soyons par principe opposés aux demandes de rapport- c'est une coutume dans cet hémicycle -, l'article 3 me semble également important. À la douleur personnelle s'ajoutent en effet trop souvent des contraintes financières, professionnelles et sociales, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Enfin, je tiens à remercier nos collègues du groupe Union Centriste d'avoir inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour des travaux de notre assemblée. Certes, ce texte comprend des dispositions qui relèvent du domaine réglementaire.

des familles. C'est pourquoi le groupe du RDSE apportera bien évidemment son soutien à ce texte, qui constitue une avancée et permettra une meilleure prise en charge et une meilleure inclusion des enfants souffrant de pathologies chroniques ou de cancers.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en France, le nombre d'enfants atteints de maladies chroniques, c'est-à-dire de maladies de longue durée, évolutives, ayant un retentissement sur la vie quotidienne, augmente régulièrement. Ainsi, depuis vingt ans, le diabète de type 1 progresse de 3 % à 4 % par an et apparaît de plus en plus précocement, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. De même, chaque année, 2 500 enfants et adolescents se voient diagnostiquer un cancer. Le nombre de ces cancers augmente de 1 % à 2 % par an en Europe depuis trente ans. À l'annonce de la maladie, c'est toute la vie de la famille qui est bouleversée.

Tout récemment, cela a été rappelé, notre assemblée a été amenée à discuter de la proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu. Promulguée le 16 novembre 2021, cette loi permet le renouvellement de la durée du congé de présence parentale, qui peut être portée à 620 jours sociale pour 2022 revoit à la hausse le montant de l'allocation journalière de présence parentale en prévoyant sa revalorisation annuelle par référence au SMIC.

L'article 1 crée un nouveau droit à congé pour événements familiaux lors de l'annonce de la survenue d'une pathologie chronique. Il s'agit là d'une mesure d'urgence, un amortisseur face au choc de l'annonce, qui consacre une certaine égalité face aux employeurs. Ce congé d'une durée de deux jours permettrait aux parents de s'occuper de leur enfant sans que cette absence soit décomptée de leurs congés payés ni qu'ils perdent une partie de leur salaire, comme c'est le cas avec les congés pour garde d'enfant malade. Si cette mesure représente une avancée par rapport au droit existant, la durée de ce congé nous paraît bien faible face aux bouleversements et aux difficultés auxquels ces parents sont confrontés.

L'article 2 relève pour nous davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif. Il instaure une réunion obligatoire sur les modalités du projet d'accueil individualisé et

Cependant, pour les parents, confier leur enfant à un tiers peut susciter de nombreuses interrogations, souvent même du stress. Cette réunion entre l'équipe encadrante et les familles pour organiser le retour de l'enfant est donc primordiale. Certes, les possibilités de concertation et de coordination existent déjà dans les faits. Cependant, dans la pratique, les entretiens ont souvent lieu trop tard. L'enjeu de cet article était donc de réduire le délai de tenue de cette réunion destinée à permettre l'adaptation de la scolarité de l'élève

ce délai obligatoire. Nous sommes également favorables à la mise en place de formations spécifiques pour les enseignants, les éducateurs sportifs et l'ensemble des équipes, ainsi qu'à la sensibilisation des futurs enseignants aux problématiques liées aux pathologies chroniques et aux cancers. L'article 3 prévoit la communication du PAI au centre d'examen, celui-ci pouvant indiquer « si la présence d'un professionnel de santé dans le centre d'examen est souhaitable lors de ces épreuves La présence d'un professionnel de santé dans un centre d'examen relève pour nous de l'incantatoire. En effet, la médecine scolaire est exsangue. En 2016, le taux moyen d'encadrement variait de 2 000 à 46 000 élèves par médecin et certains départements n'avaient même plus de médecin de secteur. À titre d'exemple, on compte un médecin scolaire pour 3 000 élèves à Paris et un médecin pour 99 000 en Dordogne, alors qu'il faudrait un médecin pour 5 000 élèves, voire pour 3 000 en zone difficile. Depuis 2013, la moitié des postes offerts au concours- cinquante par an -ne sont pas choisis et demeurent vacants. La profession de médecin scolaire risque de s'éteindre.

Alors que nous appelons tous de nos voeux une école plus inclusive, nous ne nous donnons pas les moyens d'y parvenir. Nous le déplorons. Nous le voyons, cette proposition de loi est de portée modeste, son sujet ainsi que sa disposition principale, à savoir l'instauration d'un congé de deux jours payé par l'employeur à l'annonce d'une telle maladie, oblige. Reste que, avec la stratégie des petits pas, on est toujours loin d'un statut de parent accompagnant.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui concerne des milliers d'enfants et de familles. L'objectif, sur cet hémicycle, est simple : il s'agit d'améliorer et de faciliter l'accompagnement des enfants atteints d'une pathologie chronique ou d'un cancer. fait écho, entre autres, à une autre proposition de loi que le Sénat a examinée au mois d'octobre dernier, promulguée depuis, visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu. Les débats parlementaires réguliers, qui ont donné lieu à des avancées concrètes, démontrent la volonté du législateur de permettre aux parents d'accompagner leur enfant dans les meilleures conditions possible. Il s'agit, nous le savons, d'un sujet douloureux- je pense notamment au cancer. Il est douloureux avant tout pour l'enfant, qui doit apprendre à vivre avec la maladie et son traitement douloureux aussi pour les parents, pour qui le diagnostic d'une pathologie chronique ou d'un cancer est un choc et nécessite une disponibilité immédiate. Cette proposition de loi entend envoyer un signal fort, que nous partageons. Votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, elle permettra de répondre en partie aux attentes et aux préoccupations des enfants et de leur famille. Ce texte instaure notamment un congé spécifique de deux jours pour les parents lors de l'annonce d'une pathologie chronique ou d'un cancer, sur le modèle de ce qui est prévu dans le code du travail pour l'annonce d'un handicap. Il s'agit là d'une mesure de sécurité pour les parents qui font face à l'urgence et qui se doivent d'être auprès de leur enfant. texte instaure également une réunion de l'équipe éducative au plus tard dans les trois semaines qui suivent l'entrée dans l'établissement de l'enfant malade, avec l'accord des parents, afin de favoriser une meilleure coordination. Cette disposition nous semble essentielle, car un enfant est aussi un élève. Le rôle de l'école de la République est justement de lui offrir une scolarité normale, quelle que soit sa situation. d'ailleurs ici le travail des enseignants et des personnels de l'éducation nationale, mobilisés pour garantir une continuité éducative à chacun d'entre eux. Un certain nombre de dispositifs existent pour permettre à l'enfant de retourner à l'école, lorsque cela est possible, dans les meilleures conditions. Je pense notamment au projet d'accueil individualisé, destiné aux enfants qui ont des problèmes de santé nécessitant des aménagements. Ce PAI vise précisément à leur offrir un accueil et un accompagnement individualisé. Il subsiste néanmoins des situations qui créent un sentiment de « double peine », lorsque l'enfant est exclu de certaines activités auxquelles tous ses autres camarades ont droit dans le cadre scolaire ou périscolaire, freinant ainsi sa socialisation, son développement et son émancipation. Les conséquences de la pathologie de l'enfant sur sa scolarité étant parfois méconnues, la réunion de l'équipe éducative prévue dans le texte constitue une avancée notable : elle permettra notamment aux enseignants de mieux appréhender les besoins de l'enfant, grâce également à une documentation spécialisée. Enfin, ce texte rend possible la présence d'un médecin ou d'un infirmier scolaire dans les centres d'examens durant les épreuves. Cette présence rassurera l'enfant, qui pourra passer son examen en étant sécurisé, mais aussi les parents, profondément attachés à sa réussite éducative. Les membres du groupe RDPI partagent pleinement les objectifs de cette proposition de loi. Les problématiques qu'elle traite font partie du quotidien de milliers d'enfants et de familles. Ils ont la conviction qu'elle apporte des réponses concrètes à leurs préoccupations. C'est pourquoi nous voterons avec enthousiasme cette proposition de loi. Madame

président de la commission de l'économie sectorielle et de la politique économique, président du groupe d'amitié Géorgie-France. Cette délégation est accompagnée par nos collègues Alain Houpert, président du groupe interparlementaire d'amitié France-Caucase, et Philippe Tabarot, président délégué pour la Géorgie, ainsi que par son excellence Mme Tea Katukia, ambassadeur de Géorgie en France. La délégation effectue une visite de travail en France sur les questions européennes et économiques, notamment le tourisme et la situation des entreprises en cette période de crise sanitaire. Plusieurs réunions sont organisées aujourd'hui et demain au Sénat avec la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, la commission des affaires européennes, la délégation aux entreprises et le groupe d'amitié. Les liens avec la France sont anciens, nos relations avec la Géorgie sont étroites depuis l'indépendance retrouvée en 1991 et la coopération interparlementaire est soutenue. La Géorgie poursuit ses réformes dans un contexte parfois difficile. Elle peut cependant s'appuyer sur ses atouts : riche de sa longue histoire, de son patrimoine naturel et monumental, elle est surtout forte de son peuple, qui a marqué à diverses reprises son attachement à la démocratie et à l'État de droit. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à M. David Songhulashvili et à sa délégation la plus cordiale bienvenue au Sénat français. Nous reprenons

Son médecin traitant ne répond pas, ses parents l'emmènent aux urgences de l'hôpital. Le personnel soignant les accueille, pose les questions d'usage, mais il faut faire vite, car Paul a de plus en plus mal. Des examens sont effectués. Une masse sombre est très vite détectée au niveau des reins. Ce n'est pas bon signe, des examens complémentaires sont nécessaires. Paul passe la nuit à l'hôpital, ses parents trouvent une place à ses côtés. Au petit matin, la nouvelle tombe : on diagnostique chez Paul un néphroblastome, qui apparaît chez l'enfant de moins de 5 ans et représente entre 5 % et 14 % de l'ensemble des cancers de l'enfant. En une nuit, la vie de cette famille a basculé. Elle sera désormais rythmée par ce combat, que tous ses membres vont entreprendre ensemble : tout mettre en oeuvre pour que Paul s'en sorte. Ces parents sont confrontés à une expérience que 2 500 autres couples de parents vivent chaque année en France et à laquelle ils ne sont pas préparés. L'article 1 de la proposition de loi discutée aujourd'hui permettrait aux parents de Paul de bénéficier d'au moins deux jours de congés. reconnaît à ces parents et à ceux d'enfants malades chroniques les mêmes droits que ceux dont l'enfant est porteur d'un handicap. Ces deux jours de congés seront les bienvenus et seront largement utilisés pour essayer de comprendre dans quelle nouvelle vie ils viennent de basculer, comment réorganiser tout leur quotidien pour que Paul ait toutes les chances de s'en sortir. vue administratif, beaucoup de points sont déjà prévus et le dossier qui sera remis aux parents liste toutes les démarches administratives qu'ils devront entreprendre. Le cancer ou les maladies chroniques faisant partie des affections de longue durée, les frais de santé et de transport sanitaire seront couverts par la sécurité sociale, ce qui est un soulagement pour les proches. toutefois à régler tous les autres détails de la vie pratique : se libérer du temps pour faire face au protocole thérapeutique prévu, mais aussi à tous les imprévus, et veiller à ce que la vie quotidienne puisse continuer, presque comme avant. Le code du travail permet de garantir l'emploi et le salaire du salarié pendant le congé de présence parentale, lequel peut durer jusqu'à 310 jours renouvelables. Ce congé pourra être complété par un congé pour enfant malade d'un mois par an. Un parent indemnisé par Pôle emploi sera lui aussi protégé par cette disposition. Le salaire non perçu pendant cette durée sera compensé partiellement par les allocations journalières de présence parentale, mais celles-ci sont plafonnées à un peu moins de 1 000 euros par mois par personne. Comment faire face à l'ensemble des coûts induits par la maladie de son enfant avec des revenus réduits- aides à domicile, gardes d'enfants, matériels supplémentaires, transports ?

Or ces maladies chroniques ou cancers de l'enfant sont des bouleversements majeurs dans la vie des parents, qui ont alors un besoin encore plus fort de souplesse et d'accompagnement. Il est indispensable qu'un statut mieux adapté soit mis en place le temps de la maladie de l'enfant

Ce retour à la vie « normale », même adaptée, est ce dont l'enfant malade a besoin. Ce sera aussi pour lui un gage de guérison plus rapide, une aide psychologique appréciable. Cette coordination entre professionnels et parents est une étape indispensable dans la nouvelle vie de l'enfant. Je me félicite que cette disposition soit incluse dans la proposition de loi que nous examinons.

Cette concertation, qui sera évolutive dans le temps et dans la forme, permettra de réadapter le protocole de prise en charge scolaire en fonction de l'évolution de la maladie et de ses manifestations. Cette proposition de loi reconnaît certains effets de la survenue de la maladie chronique ou du cancer sur l'enfant et ses parents et le bouleversement qui leur est infligé. Elle acte la nécessaire prise en charge de l'enfant par l'établissement scolaire qu'il fréquente.

et non plus obligatoire, comme cela était initialement prévu, d'un médecin ou d'un infirmier scolaire dans chaque centre d'examen durant les épreuves. Si l'ambition initiale est assez amoindrie, la raison en est très certainement l'impossibilité d'assurer l'effectivité

soient multipliés alors même que le nombre de médecins scolaires est en diminution constante : il est passé de 1 400 en 2006 à 990 seulement en 2017. La baisse des moyens alloués se cumule avec la médiocre attractivité de cette profession, due à l'absence de reconnaissance, y compris salariale, de cette spécialisation.

Le taux de visite pour les élèves de 6 ans varie selon les lieux et les départements de 0 % à 90 %. La qualité et l'égalité des soins en milieu scolaire sont clairement bafouées,

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Union Centriste, de la proposition de loi tendant à favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l'activité agricole et l'environnement, présentée par M. Pierre Louault et plusieurs de ses collègues

Un couple de jeunes agriculteurs ayant un enfant handicapé doit agrandir sa maison de plain-pied. Malheureusement, l'extension n'est possible que sur un terrain classé agricole : le permis de construire lui est refusé.

grand projet de loi. Aujourd'hui, nous allons creuser ce sujet, c'était une nécessité après la loi Climat. Souvent, nous ne traitons d'urbanisme que dans le cadre de projets de loi,

Nul besoin de vous rappeler le contexte particulier dans lequel a été conçu et présenté ce texte, dans une période marquée par le mouvement des gilets jaunes, par l'adoption de la loi portant lutte par la dynamique de retour vers la campagne de nombreux citadins danse le contexte de la crise sanitaire et économique. Les élus des zones rurales sont aujourd'hui soumis à des injonctions contradictoires, parfois inextricables enrayer le déclin démographique et économique de territoires ruraux qui, selon l'Insee, restent en moyenne plus touchés par la désindustrialisation, la précarité, la déprise agricole ou le vieillissement que le reste du pays ; lutter ainsi contre la « périphérisation » de milliers de communes et de leurs habitants ; mais aussi assurer l'avenir du secteur agricole français et mieux protéger nos sols de l'artificialisation. Les débats sur le projet de loi Climat et résilience l'ont montré : ces exigences multiples sont parfois difficiles à concilier et il n'est pas aisé de trouver un bon équilibre. Ce texte, inscrit à l'ordre du jour de nos travaux par le groupe Union Centriste, a le grand mérite de soulever une question trop souvent éludée par le Gouvernement : notre droit de l'urbanisme, pensé et conçu avant tout pour les territoires urbains et dynamiques, voire pour les zones tendues, est-il adapté aux enjeux de la ruralité ? L'une des problématiques principales de ces territoires est la dégradation de l'habitat, faute d'occupants et surtout de moyens. Dans la « diagonale du vide », 100 000 logements deviennent vacants chaque année. revient pas tant à la faiblesse de la demande qu'au manque de rénovations. Le coût de la modernisation est souvent prohibitif, mais les règles d'urbanisme, notamment de changement de destination, sont aussi parfois un obstacle. Nombre de maires déplorent que des familles renoncent à s'installer faute de trouver un logement adéquat ou d'obtenir un permis de construire. Nos nombreuses auditions ont démontré que certaines règles d'urbanisme, pertinentes pour les zones urbaines, représentent des verrous excessifs pour les petites communes rurales. Les communes dont le territoire est à dominante agricole ou naturelle ont structurellement moins de droits à construire que les communes plus urbanisées, ce qui contribue à geler leur développement.

Les propositions formulées dans ce texte apportent des pistes de réponse pour adapter le droit et lever certains verrous. Notre commission a pleinement soutenu cette démarche, qui répond à un réel besoin, dans une logique de plus grande équité entre les territoires et de vivre ensemble.

le zonage des ZRR, principalement fiscal, nous est apparu à la fois trop large- il concerne près de la moitié des communes françaises, territoires aux réalités diverses -et trop mouvant pour servir de base à des mesures spécifiques d'urbanisme. Pour refléter ce changement de ciblage, nous avons modifié l'intitulé de la proposition de loi. Ensuite, nous avons souhaité introduire une dose de territorialisation dans la politique de revitalisation rurale. En nous inspirant du dispositif dit « Pinel breton », nous proposons aux territoires eux-mêmes d'affiner le ciblage. Les intercommunalités participeront à la définition du champ d'application des dérogations d'urbanisme et des dispositifs d'aides fiscales. Les élus locaux sont ceux qui connaissent le mieux les besoins réels de leurs territoires : il faut améliorer le dialogue à l'échelon local et permettre une plus grande différenciation. nous avons souhaité soutenir l'effort de réhabilitation et de modernisation du parc de logements, car la construction nouvelle n'est pas la solution à tout. Plutôt que d'étendre l'ensemble du dispositif Pinel, qui, aujourd'hui, vise principalement le logement collectif neuf, nous avons souhaité mieux mobiliser le Denormandie pour la réhabilitation de logements anciens. Nous l'avons donc prolongé jusqu'à 2025 et en avons ouvert le bénéfice aux petites communes rurales, qui en sont à ce jour exclues. Enfin, il nous a paru nécessaire de renforcer l'encadrement de certaines mesures pour en garantir l'efficacité et l'acceptabilité. Par exemple, nous avons recentré les assouplissements en matière de constructibilité

contribuera à une meilleure lisibilité de leurs décisions. Mes chers collègues, cette proposition de loi apporte des réponses concrètes, ciblées et équilibrées au constat que nous faisons tous : il est nécessaire d'accroître les efforts de revitalisation rurale. Elle s'attelle- enfin ! -à un sujet trop souvent éludé par le Gouvernement, bien que crucial pour près de la moitié des communes françaises : comment réconcilier droit de l'urbanisme et développement rural ? J'émets donc le souhait que ce texte à la fois lucide et constructif

alors même que l'offre de nouveaux logements n'y suit pas. Face à ce constat, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Tout d'abord, nous avons créé des contrats de relance du logement dans chaque territoire tendu, financés à hauteur de 175 millions d'euros par le plan de relance. Ensuite, nous avons conclu un protocole ambitieux visant à contractualiser

pendant dix ans pour les logements sociaux agréés en 2021. Nous avons aussi choisi de porter le fonds pour le recyclage des friches de 300 à 650 millions d'euros pour 2021 et de le pérenniser afin de faciliter la mobilisation de foncier déjà artificialisé. Ces outils

Afin de construire mieux et de façon plus raisonnée, de préserver nos sols agricoles, nos espaces naturels et nos paysages, nous avons fait évoluer les normes d'urbanisme. Malgré la prise de conscience de la nécessité de préserver ces sols, le rythme d'artificialisation

comme les matériaux biosourcés. C'est d'ailleurs un des sujets phares des Assises de la forêt et du bois, que je mène actuellement avec Julien Denormandie. Il s'agit d'une activité très structurante pour nos territoires.

Pour assurer une protection effective de nos sols, de nos terres agricoles et forestières, et garantir un aménagement raisonné, nous avons procédé à une évolution majeure du code de l'urbanisme en y introduisant la notion de lutte contre l'artificialisation des sols, définie par la loi Climat et résilience du 22 août 2021.

nécessite, ou encore à la possibilité d'y construire, dans un cadre précis, tout en veillant à la préservation des terres agricoles. Il faut le redire

L'article 3 prévoit de prendre en compte la spécificité des territoires ruraux dans les documents annexes des SCoT pour l'analyse de la consommation d'espace. Il me semble déjà satisfait par l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, tel qu'il a été modifié par la loi Climat et résilience.

... L'article 5 permettrait de construire un logement sur une exploitation agricole en s'affranchissant de la prise en compte du zonage agricole et du type d'activité de l'exploitation. J'y suis également défavorable.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi n'est pas la première initiative visant à simplifier le droit de l'urbanisme. Le Sénat appelle depuis plusieurs années à desserrer l'étau normatif sur la construction en milieu rural.

Si nous sommes si nombreux depuis tant d'années à considérer que le droit de l'urbanisme n'est pas adapté aux zones rurales, qu'il paralyse le développement économique, qu'il empêche la conservation des emplois et donc des habitants,

est le fait de 10 % des communes, en particulier des métropoles. Les PLU des communes rurales se trouvent amputés de 60 % de surfaces constructibles. Vous avez affirmé à l'instant, madame la secrétaire d'État, que les communes rurales pourront continuer à délivrer des permis de construire.

chose ! Nous affirmons que les communes rurales sont gérées par des maires réfléchis, qui veulent prendre leurs responsabilités, avec liberté. Les maires ruraux sont les premiers protecteurs de la biodiversité J'évoquerai surtout l'hypocrisie de certaines dispositions du code de l'urbanisme, dont on nous dit qu'elles traduisent une préoccupation constante de préserver l'environnement. Puisqu'on ne peut pas, ou qu'on ne veut pas, rationaliser l'utilisation des sols autour des grandes métropoles, je ne reviendrai pas sur la question du « dimensionnement » de l'urbanisation. Les territoires ruraux deviennent les victimes expiatoires de notre impuissance ! La même hypocrisie règne s'agissant des éoliennes et des documents d'urbanisme. On demande aux élus de se justifier lorsqu'ils souhaitent geler certaines zones du territoire face au développement éolien. D'un côté, on demande aux élus de justifier la constructibilité d'un abri de jardin de 15 mètres carrés dans leur PLU

À défaut d'une révolution, j'en appelle surtout à des ajustements pour assurer un développement minimal dans les territoires ruraux, développement théoriquement assuré par la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre en son article 8 la liberté de choisir son domicile. Je ne me fais pourtant pas d'illusions, le Gouvernement ne sera pas particulièrement bienveillant. Si le Gouvernement est hostile aux initiatives comme celle-ci visant à libérer la construction en milieu rural, il n'a qu'à prendre ses responsabilités en matière de rénovation énergétique.

Assurément, cette proposition de loi va dans le bon sens. Certes, elle n'est pas parfaite, ses effets mettront un peu de temps à se matérialiser, mais elle constitue une des réponses que nous devions apporter. Notre groupe votera donc cette proposition de loi. Nous espérons également que notre groupe sera en mesure, malgré un calendrier législatif contraint, de proposer de nouvelles dispositions afin de redonner aux élus locaux une véritable autonomie et des moyens pour se développer. Il s'agit de redonner aux maires du pouvoir de décision

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord quelques remarques générales sur la philosophie même de cette proposition de loi. Nous soutenons, bien évidemment, les objectifs de revitalisation des territoires ruraux peu denses, car il est primordial d'engager le désengorgement de nos métropoles et de réinvestir nos petites villes, ainsi que nos campagnes. Nous nous retrouvons moins sur le raisonnement qui induit que la revitalisation d'un territoire passe nécessairement par la construction de bâtiments neufs. Nous pensons que la revitalisation passe davantage par le déploiement de services publics, de commerces de proximité et, bien sûr, par la réhabilitation du bâti.

l'objectif de diminution de moitié de l'artificialisation des sols à l'horizon de 2030. C'est en ce sens que nous avons déposé un amendement de suppression de l'article 2. L'assouplissement des règles de constructibilité sur l'ensemble des terrains agricoles en continuité d'un espace urbanisé, comme le prévoit ce texte, risque de favoriser le mitage, le mitage, si coûteux pour les communes et les terres agricoles. La problématique vaut également pour l'assouplissement, qui est étendu à toute l'exploitation et plus seulement au périmètre regroupant les bâtiments de la ferme.

Par ailleurs, nous souhaitons,, réintroduire l'avis conforme des CDPENAF dans les différents cas où il est mentionné. Cette commission est un outil utile dans la lutte contre l'artificialisation des terres et subit de nombreux affaiblissements alors qu'elle devrait être renforcée. Le travail au sein de ces commissions permet d'améliorer les projets et donc d'éviter des refus précoces ou des contentieux chronophages et coûteux pour les communes. Quant aux changements de destination des bâtiments agricoles prévus également à cet article, ils doivent être encadrés strictement. Si le développement de l'habitat des agriculteurs est déjà possible dans le cadre législatif actuel, nous sommes bien conscients que certains verrous juridiques peuvent perdurer, notamment au moment de l'installation. Des solutions sont possibles pour améliorer l'accès au logement pour les agriculteurs sans ouvrir la porte à une artificialisation trop peu maîtrisée des sols. Un rapport du Gouvernement sur les initiatives actuelles permettrait d'identifier les pratiques mises en oeuvre sur le terrain et les politiques publiques efficaces pour les soutenir. C'est ce que nous proposerons à l'article 5. Enfin, l'article 6 nous paraît largement inutile, le droit existant, la reconnaissance de la « pré-occupation », étant déjà protecteur en la matière, comme le souligne le Conseil d'État. Il semble donc nécessaire de ne pas modifier les équilibres existants pour ne pas heurter le principe du droit d'agir en responsabilité et, plus généralement, du droit au recours effectif. C'est pourquoi nous proposerons la suppression En conclusion, cette proposition de loi ne nous paraît pas pertinente pour répondre aux enjeux de revitalisation des territoires ruraux, la priorité étant, pour notre groupe, la réhabilitation des logements vacants, la présence des services publics, le maintien de l'emploi agricole et paysan.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi de nos collègues du groupe Union Centriste, qui vise à favoriser l'habitat en zone rurale tout en protégeant l'activité agricole et l'environnement. Nous partageons clairement ses considérants et son objectif : permettre aux communes de revitaliser leur territoire. Il est vrai que le code de l'urbanisme a évolué ces dernières années afin de réduire l'artificialisation des sols et de limiter l'étalement urbain. Pourtant, cet objectif, juste et légitime, a malheureusement conduit à une quasi-interdiction des constructions en zone rurale. En effet, le code de l'urbanisme impose aux collectivités de fixer des objectifs en fonction de l'évolution démographique d'un territoire cours des années précédentes. Il en résulte que les petites communes rurales, dont la population évolue peu, ne peuvent plus délivrer de permis de construire. C'est une forme de double peine puisqu'à la déprise démographique s'ajoute l'impossibilité d'accueillir de nouveaux habitants. Cette situation est inacceptable alors que la crise sanitaire a suscité un réel engouement pour la ruralité. Cette proposition de loi est donc intéressante, d'autant que son passage en commission

reste incertain. Elle vise désormais l'ensemble des petites communes, plus particulièrement celles qui ne disposent pas de plan local d'urbanisme et qui sont donc soumises La proposition de loi permet la construction en continuité urbaine des bourgs et hameaux, ainsi qu'un changement de destination de certains bâtiments, notamment au sein des exploitations agricoles. Ces facultés ont été recentrées sur la seule nécessité de produire des logements ou des hébergements, et ce uniquement dans la continuité de l'espace déjà urbanisé à la date de la présente proposition de loi. Cet équilibre nous semble pertinent pour éviter un mitage trop important des terres agricoles.

est également la conséquence d'une perte majeure d'ingénierie au sein des collectivités en zone rurale. La suppression de l'assistance technique de l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (Atésat) et la redéfinition de l'application du régime des autorisations du droit des sols (ADS) ont conduit à de grandes disparités territoriales.

Par ailleurs, les situations de blocage peuvent également être liées à la création d'intercommunalités forcées, les plus petites communes se trouvant dans un rapport de force ne leur permettant pas de partager leurs projets urbains et une vision dynamique de leur territoire. Les différentes lois qui se sont succédé, telles que la loi pour l'accès au logement et un

ruraux ne suivent pas. Cette proposition de loi vise également à faciliter l'exercice des activités agricoles. Il s'agit notamment de reconnaître le droit pour chaque agriculteur de vivre sur son exploitation. C'est une idée que nous partageons. Aujourd'hui, de plus en plus de bâtiments agricoles sont en ruine sur nos territoires. C'est, de mon point de vue, une bonne chose que de permettre leur réhabilitation

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, grâce à la démarche de Pierre Louault et aux apports de Valérie Létard, que je tiens à saluer et à remercier pour leur engagement sur ce texte, la présente proposition de loi tend à donner à la ruralité les moyens de ses ambitions et de relever ses difficultés. Il n'échappe à personne que les campagnes se vident depuis plus d'un siècle, que les « places du marché » et les « rues du commerce » sont moins fréquentées, et que les bras manquent dans les fermes, quand celles-ci ne disparaissent pas. Ce tableau n'est pas nouveau, il est celui d'une France qui a passé le pas de la modernité il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Nul besoin, toutefois, de ressasser les images du passé : j'ai l'intime conviction que la ruralité regorge de ressources qui lui permettront de sortir de l'ornière. Parmi ces ressources, il y a l'habitat. Loin des prix faramineux de l'immobilier dans les métropoles, les territoires ruraux sont

Si l'exode rural se poursuit, l'exode urbain est une réalité de plus en plus tangible. Paris a ainsi perdu près de 54 000 habitants entre 2013 et 2018. Il est aujourd'hui nécessaire de donner aux territoires ruraux les moyens de leurs ambitions en matière de logement et de valorisation du patrimoine,

Il ne s'agit pas de discuter ces objectifs, car freiner la consommation du foncier agricole est aujourd'hui un enjeu stratégique national. Il s'agit plutôt de montrer que les territoires ruraux sont pénalisés et disposent de peu de zones constructibles alors même qu'ils en ont de plus en plus besoin pour briser le cercle vicieux de la dévitalisation.

Nous nous faisons tous, mes chers collègues, les relais des difficultés que rencontrent les agriculteurs de nos départements respectifs. C'est une profession tout entière qui rencontre les mêmes difficultés économiques, administratives, climatiques ; celles-ci ont même pour effet de dissuader les plus chevronnés de poursuivre leur activité et les jeunes les plus motivés de s'installer. Notre responsabilité, en tant que législateurs, est de lever ces freins à l'installation. Je me réjouis donc que cette proposition de loi contienne des dispositions ambitieuses à ce sujet. proposition de loi en faveur du développement de l'habitat dans les zones rurales et du maintien de l'activité agricole est donc salutaire et porte sur deux socles essentiels de la revitalisation des territoires ruraux. Cette ambition a a été réaffirmée par la commission des affaires économiques, qui a su enrichir ce texte avec justesse et bon sens, par exemple en remplaçant revitalisation rurale par des mesures d'assouplissement ouvertes à l'ensemble des communes de petite taille et des mesures plus larges au bénéfice des communes peu denses en déprise démographique. Ces mesures faciliteront la transformation d'anciens corps de ferme ou de granges inoccupés en logements dans tous les territoires ruraux, sans limiter l'application d'une telle disposition à un zonage administratif spécifique. La commission a également amendé le texte initial afin de sécuriser le droit au logement des agriculteurs sur leur exploitation. Elle a confirmé son soutien aux agriculteurs en considérant que les troubles inhérents à l'activité agricole causés sur le voisinage ne sont pas considérés comme des dommages si l'activité agricole préexiste aux habitations concernées. Les coqs pourront ainsi continuer de chanter ! C'est donc en soutien à nos territoires ruraux et eu égard à la qualité de la présente proposition de loi que le groupe Union Centriste votera naturellement ce texte,

tous les observateurs s'accordent à souligner que la crise que nous traversons a eu pour conséquence un regain d'intérêt pour les territoires ruraux. Les qualités de nos territoires sont enfin connues et reconnues. Nous ne pouvons que nous en réjouir Comme le rappelait Alain Bertrand dans son rapport, nous disposons d'un potentiel de développement économique, social et écologique qu'il faut pouvoir accompagner, mais comment y arriver si nous n'avons pas la capacité d'accueillir de nouvelles populations ? C'est ce retour à la campagne que les auteurs de la présente proposition de loi entendent accompagner. L'objectif est non pas de tout déréglementer, mais de lever les verrous qui sont Assouplir, autoriser l'urbanisation et permettre les changements de destination de certains biens à des fins d'habitation dans nos zones hyper-rurales constitue une réponse adéquate. Cependant, appliquer à tous les territoires la même règle, c'est la double peine Les territoires ruraux ont subi pendant des années l'absence de véritable politique d'aménagement du territoire et un recul constant des services publics. Est-il juste aujourd'hui de leur refuser de construire au motif qu'ailleurs nous avons consommé trop d'espace ? loi ne peut pas nous priver du droit à l'accueil dont ont bénéficié pendant longtemps les métropoles et les agglomérations. Notre législation doit être adaptée. Tel est l'objectif de ce texte,

concerne l'extension du dispositif Denormandie dans l'ancien, je m'interroge sur son recentrage sur les communes rurales qui disposent d'un fort taux de vacance. À mon avis, cette disposition rate sa cible. Nous proposerons donc un amendement visant à l'étendre aux autres communes peu denses ayant un besoin de logement avéré. Pour autant, je partage l'idée que nous devons nous interroger sur ces 100 000 logements qui deviennent vacants tous les ans. C'est en traitant cette question que nous préserverons nos terres de l'artificialisation et non en mettant sous cloche les territoires peu peuplés. Certes, les dispositions du projet de loi 3DS faciliteront quelque peu l'acquisition des biens sans maître ou des biens abandonnés. Mais pour être efficace, il faut des mesures fiscales en faveur de la rénovation de l'existant. Nous savons que l'inadaptation des logements anciens aux besoins actuels et le coût de leur rénovation sont des freins à l'acquisition. Enfin, je précise que nous sommes également favorables à l'article 6 relatif aux troubles inhérents aux activités agricoles. Pour conclure, je remercie les auteurs de la proposition de loi. Le texte répond à une préoccupation constante des élus qui se démènent pour maintenir la vie dans leurs villages. Ayons toutefois toujours à l'esprit que nos difficultés ne se limitent pas à l'habitat. Nous avons également des besoins urgents en termes d'infrastructures, de services publics, de commerces de proximité, d'emplois. Toutefois, nous allons dans la bonne direction. Le groupe RDSE votera donc cette proposition de loi. Madame

j'ai le plaisir de saluer, dans la tribune d'honneur, une délégation de la Grande Assemblée nationale turque conduite par M. Mehmet Kasım Gülpinar, président du groupe d'amitié Turquie-France. Elle est accompagnée par M. Jean-Claude Requier, président du groupe d'amitié du Sénat. Après des entretiens à l'Assemblée nationale, la délégation a assisté au Sénat au colloque co-organisé par le groupe d'amitié et le comité France-Turquie sur les cent ans du traité d'Ankara. Cet accord signé, le 20 octobre 1921 par le ministre des affaires étrangères du Gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Yusuf Kemal, et l'envoyé spécial du Gouvernement français, Henri Franklin-Bouillon, mit fin immédiatement à l'état de guerre entre la France et le Gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie. La France ouvrait ainsi la voie à la reconnaissance internationale de la Turquie nouvelle du Gouvernement de M. Mustafa Kemal. La délégation turque vient d'avoir des entretiens avec le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, M. Christian Cambon, et avec le vice-président de la commission des affaires européennes du Sénat, M. André Reichardt. Cette visite renoue avec une relation essentielle pour la stabilité, la sécurité et la prospérité de nos deux pays. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à M. Mehmet Kasım Gülpinar et à sa délégation la plus cordiale bienvenue au Sénat français.

est le constat des auteurs de ce texte, auquel nous ne pouvons que souscrire. Il faut en effet trouver un équilibre entre le développement de l'habitat, des activités et des services à la population, tout en protégeant l'activité agricole et l'environnement. Je tiens d'abord à saluer le travail de la rapporteure qui, par ses propositions, a fait évoluer le texte sur deux points sur lesquels nous avions une position défavorable. Le premier point concerne le périmètre retenu, pour faciliter l'accès à l'habitat dans les territoires en déprise démographique. Ce périmètre ne nous paraissait pas pertinent pour trois raisons. Tout d'abord, parce qu'une réflexion doit être prochainement engagée pour réviser les dispositifs zonés. Ensuite, parce qu'il n'inclut pas l'ensemble des territoires ruraux. Enfin, parce que les ZRR comprennent des communes très diverses, qui ne rencontrent pas les mêmes difficultés. Nous sommes donc favorables au fait de viser les communes rurales peu denses en déprise démographique, plutôt que les ZRR.

Le deuxième point de blocage portait sur l'article 4, qui prévoyait d'appliquer le dispositif Pinel aux ZRR. Nous n'y étions pas favorables, car nous estimons, comme la rapporteure, que le dispositif Denormandie dans l'ancien, qui est un avantage fiscal en faveur de la rénovation du bâti, est plus adapté aux spécificités des territoires ruraux. Depuis le début de la pandémie, nos concitoyens ont redécouvert le potentiel offert par l'habitat en zone rurale. Afin de parvenir à un équilibre, il est donc indispensable de ne pas accentuer les inégalités territoriales.

mais pas seulement. La déprise démographique ne résulte pas uniquement d'un manque de logements ou de contraintes trop importantes en matière d'urbanisme. Permettre l'arrivée d'une nouvelle population nécessite aussi l'implantation d'activités, de services et d'infrastructures. L'objectif de la proposition de loi telle qu'elle ressort des travaux de la commission est bien d'accompagner nos territoires pour qu'ils disposent des outils nécessaires au renouvellement de leur patrimoine existant et au développement de leur attractivité. Nous sommes donc favorables à ce texte. La parole est

Pour ma part, j'en connais un certain nombre, si bien que je ne peux que porter un regard bienveillant sur cette proposition de loi. Bien ! Ce texte cible en effet un blocage que je rencontre trop souvent, d'autant que depuis la crise sanitaire les spéculations vont bon train sur une « dé-métropolisation » de la France.

Comment répondre à cette nouvelle demande ? C'est peut-être sur ce point que nous divergeons. La proposition de loi prévoit de permettre à n'importe quelle commune en déprise démographique, disposant ou non de documents d'urbanisme, de déroger au droit de l'urbanisme. Elle offre ainsi des assouplissements en matière de construction nouvelle, d'adaptation du bâti et de changement de destination, en particulier dans les zones naturelles, agricoles et forestières.

ce point. Permettez-moi néanmoins de vous faire part de mes interrogations. À mon sens, ce texte avantage en premier lieu les communes régies par le règlement national d'urbanisme. Elles sont environ 10 000, mais que va-t-on dire aux 25 000 autres, soit 70 % des communes, qui, elles, ont fait l'effort financier de réaliser un document d'urbanisme ? Contrairement aux idées reçues, toutes ne sont pas des collectivités urbaines richement dotées, loin de là que nous avons prises pour lutter contre l'artificialisation des sols, qui figurent tout de même dans une cinquantaine d'articles de la loi Climat et résilience. Rappelons que la loi a fixé un objectif national d'absence d'artificialisation nette d'ici à 2050. Dit autrement, déroger au droit de l'urbanisme, c'est favoriser le mitage par l'installation de bâtiments ou de logements dans le paysage rural, sans lien avec le schéma de cohérence territoriale et en totale contradiction avec la loi Littoral ou la loi Montagne. Enfin, dans les communes régies par le RNU, si on ne peut pas construire en dehors des espaces attribués, on peut tout à fait bâtir en fonction des besoins de la commune. Il est par exemple possible de changer la destination des bâtiments agricoles pour en faire du logement ou de construire de nouveaux bâtiments à usage d'habitation dans le périmètre de bâtiments agricoles existants. Et surtout, pour éviter la perte démographique, il est possible de construire en dehors des espaces urbanisés sur délibération motivée de la commune. Mes chers collègues, je veux que l'on puisse trouver des solutions pour nos maires qui connaissent ces difficultés, mais les dispositifs ici proposés sont disproportionnés et inéquitables pour l'ensemble de nos collectivités. Il est nécessaire de travailler avec le Gouvernement pour trouver des solutions pertinentes. Ainsi, pourquoi ne pas prévoir un dispositif d'incitation en direction des maires souhaitant réaliser un document d'urbanisme

à Murat, en 2004, le président de la République Jacques Chirac évoquait « l'attachement de notre pays à une ruralité moderne ». Je pense que c'est toujours le cas- j'ajouterai, en le paraphrasant quelque peu, à une ruralité heureuse -quand je vois l'énergie que sont prêts à déployer nos territoires les plus ruraux pour relever le défi du dynamisme et de l'attractivité. Cette proposition de loi est importante, car elle traduit une volonté de permettre à nos territoires les plus ruraux de faire face aux défis actuels en matière d'urbanisme. Je tiens à saluer notre collègue Pierre Louault pour son engagement, ainsi que la commission des affaires économiques, dont le travail a permis d'affiner ce texte. Depuis quelques années, les territoires ruraux retrouvent une certaine vitalité et sont de plus en plus attractifs.

Les citoyens qui y habitent ont les ressources pour faire évoluer notre pays et ses territoires. Ils sont attachés au développement des bassins de vie et souhaitent y impulser un nouveau dynamisme. Néanmoins, nous faisons face au problème majeur de l'artificialisation des sols. Notre pays a amorcé une transition nécessaire dans bien des domaines. Nous ne nions absolument pas l'importance de freiner la consommation de nos sols, mais force est de constater qu'une

C'est apporter de l'équilibre et de la flexibilité au rythme de freinage. Enfin, ce n'est que justice pour des territoires qui sont confrontés à un paradoxe : un regain d'attractivité et une impossibilité d'accueil. Pour redonner du dynamisme à notre hyper-ruralité, il faut rompre ce cercle vicieux.

qui nous est aujourd'hui soumis. Cette proposition de loi s'appuie sur un constat simple : le déclin démographique de nos villages ruraux. Ce constat, nous le partageons. Il repose d'ailleurs sur une donnée objective, qui, pour notre groupe, est essentielle notre groupe, est essentielle : la part de logements vacants est bien plus importante dans nos communes rurales que dans le reste de la France. L'attractivité naturelle de nos villages n'est pas en cause. Il nous appartient donc d'apporter des réponses politiques à ce phénomène.

L'une des façons de préserver des services de proximité et des services publics dans nos villages, c'est d'y maintenir et d'y attirer les populations. Pour ce faire, nous devons adapter nos règles urbanistiques règles urbanistiques qui, comme leur nom semble l'indiquer, sont peut-être parfois un peu trop urbaines et éloignées des réalités et des spécificités de nos territoires ruraux. Clairement, il nous faut porter une ambition de revitalisation rurale. Cette ambition ne doit pas pour autant nous faire oublier nos objectifs de préservation de l'environnement et de sauvegarde des terres agricoles. Alors oui, il arrive que des exigences soient pertinentes et légitimes, tout en étant potentiellement contradictoires dans leur application. Dans ce genre de situation, il faut savoir donner des marges de manoeuvre et un pouvoir de décision et d'arbitrage aux élus locaux. Tel est le sens de cette proposition de loi, à laquelle nous souscrivons.

Pour autant, nous émettons une réserve qui a son importance. J'ai déjà évoqué la question centrale de la vacance des logements. Dans le cadre de notre objectif commun, la lutte contre cette vacance aurait dû être la première des priorités. La réappropriation du bâti existant permettrait de sauver le patrimoine qui fait le charme de nos communes et de renforcer leur attractivité tout en limitant l'habitat diffus et ses conséquences. Bien Bien sûr, un tel projet nécessiterait un plan massif d'accompagnement des maires désireux de s'engager dans cette démarche. À l'inverse, si nous faisons des constructions nouvelles une priorité, le risque est d'augmenter la vacance, d'accroître le délabrement du bâti existant et, de fait, de réduire l'attractivité et la vitalité de nos communes, contrairement à notre ambition initiale.

51 % des ruraux estiment que le monde rural est abandonné, notamment en raison des problèmes d'accessibilité aux services publics, de la fracture médicale et numérique, des problèmes de mobilité et d'autres causes qui entretiennent un sentiment d'abandon. Ces espaces relégués

en faveur de ces territoires fragiles. Il tend à étendre la portée de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme à l'ensemble des territoires caractérisés par des handicaps géographiques, économiques et sociaux clairement identifiés par l'Insee et qui bénéficient à ce titre de politiques renforcées et différenciées de développement allant au-delà des dispositifs fiscaux attachés à la zone de revitalisation rurale, dont la portée n'est à ce jour pas garantie au-delà de 2022.

Il faut arrêter d'accentuer les ruptures territoriales. Au contraire, il faut engager une profonde évolution de notre rapport aux territoires, dans un objectif de préservation et de cohésion. Aussi, il nous semble important de compléter l'article 1 qui cible les seules

Merci

par cohérence avec notre position en commission et à viser l'ensemble de la ruralité. Deuxièmement, il tend à compléter les grands objectifs figurant déjà dans le code de l'urbanisme afin de mieux mettre en valeur et de renforcer les objectifs liés à la ruralité, dans le prolongement de ce qu'a voté le Sénat, sur l'initiative de notre commission, dans la loi

conduirait à menacer l'équilibre, que nous souhaitons préserver, entre les populations qui résident dans les zones urbaines et les populations rurales. D'ailleurs, les dispositions de l'article L. 101-2 sont d'ordre général : elles s'imposent aux documents de planification.

M. Daniel Salmon. Nous proposons la suppression de l'article 2 pour plusieurs raisons. L'assouplissement des règles de constructibilité applicables à l'ensemble des terrains agricoles en continuité d'un espace urbanisé prévu par cet article risque de favoriser le mitage et donc l'artificialisation des sols. assouplissement est également étendu à toute l'exploitation, et plus seulement au périmètre regroupant les bâtiments de la ferme. Ces dispositions vont à l'encontre de nos objectifs de protection des espaces agricoles. Le « changement de destination des constructions existantes aux fins de création de logement et d'hébergement » est un périmètre bien trop large. Il existe un risque réel de transformer n'importe quel bâtiment agricole en habitation, même si son usage initial en était très éloigné. Le terme « constructions » est très vague.

doit se faire de façon parcimonieuse et ne doit pas mettre à mal la préservation des sols et de la biodiversité. Certains ici- très rares, je le concède -rêvent encore du pavillon

Les dispositions applicables au RNU prévoient actuellement des possibilités de construction en dehors des parties urbanisées de la commune. Elles permettent par exemple de faciliter « le changement de destination, [ ...] l'extension des constructions existantes ou [encore] la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole ». Ces dispositions, nous les avons travaillées collectivement au cours des dernières années, pour arriver à un juste équilibre entre, d'une part, la protection du foncier agricole

ni de continuité du bâti. Au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer cette modification, qui ne nous paraît pas souhaitable, car, selon la taille des terrains concernés, elle risque de favoriser la création d'habitats diffus à proximité d'activités agricoles. Nous en connaissons tant les inconvénients au regard de l'environnement que les coûts pour la collectivité.

La CDPENAF est un outil de lutte contre l'artificialisation des terres naturelles, agricoles et forestières. Elle est très utile ; ce texte l'affaiblit, alors qu'elle mériterait au contraire d'être renforcée.

maintenue, elle devrait être assujettie à l'avis conforme de la CDPENAF, au même titre que les autorisations de construction déjà visées par le code de l'urbanisme, motivées par la volonté d'éviter la diminution de la population communale et à condition que les constructions envisagées ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Bouad. La présente proposition de loi permet aux règlements de PLU de prévoir, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, la possibilité de constructions nouvelles sur l'ensemble des terrains sur lesquels sont situés les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole. Dans la logique de nos amendements précédents, nous proposons de supprimer ces nouvelles ouvertures à la construction. En effet, sans encadrement plus précis, cette possibilité risque d'être la source d'un habitat dispersé, auquel, vous le savez, nous ne sommes pas favorables.

il est aujourd'hui possible de construire sur une ancienne ferme, mais uniquement dans le « périmètre bâti », notion que les préfets et les juges interprètent, de façon très restrictive, comme désignant l'intérieur de la zone délimitée par les contours extérieurs des bâtiments. En conséquence, il est souvent refusé, par exemple, de construire un petit logement agricole sur la grande cour arrière d'un ancien corps de ferme, si les bâtiments anciens de la ferme sont très rapprochés. Or, dans cet exemple, on ne parle pas de terres cultivées ni même végétalisées. L'évolution vise donc à permettre une petite souplesse supplémentaire, afin de ne pas se limiter au

assez simple. Il est effectivement possible de construire des bâtiments d'habitation à l'intérieur du périmètre d'une installation, mais l'extension de cette possibilité à l'ensemble du terrain, parfois vaste, de l'exploitation conduirait très clairement à un mitage. De la même façon, il me semble souhaitable d'imposer la délivrance de l'autorisation sollicitée à un avis conforme de la CDPENAF, ce qui nous permet de mieux contrôler les constructions et leurs principaux impacts négatifs éventuels.

La règle de « constructibilité limitée » applicable dans les communes soumises au RNU limite les possibilités de délivrer des autorisations de construire aux seules parties urbanisées de la commune. Des exceptions prévues dans le code de l'urbanisme permettent de délivrer des autorisations, notamment pour des « changements de destination » ou une « extension des constructions existantes ». Les services instructeurs considèrent généralement que, lorsque l'extension dépasse 30 de la surface d'origine, l'opération est requalifiée en nouvelle construction. La demande de permis de construire est alors rejetée, en application de l'interdiction des constructions nouvelles en dehors des parties urbanisées de la commune, ce qui n'a pas de sens. Pour apporter de la souplesse à la notion d'« extension des constructions existantes », nous proposons, les projets d'extension « eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur dimension n'excédant pas les deux tiers de la construction d'origine ». Notre objectif est bien la reconquête du bâti des centres-bourgs et des centres de village, l'idée étant de valoriser et de favoriser la réappropriation du bâti existant dans les petites communes.

des fermes existantes. La loi ne fixe pas de limite chiffrée à cette extension tant que cette dernière ne constitue pas une nouvelle construction. C'est une bonne chose que la loi ne fixe pas de seuil arbitraire, car il est parfois nécessaire, pour moderniser un vieux bâtiment agricole ou rénover un corps de ferme, d'agrandir Cela facilite le réemploi de ces derniers et la revitalisation des zones rurales. Inscrire dans la loi un plafond chiffré serait plus restrictif que le droit actuel et irait à l'encontre de notre objectif, qui est de faciliter la modernisation du bâti existant. D'ailleurs, dans l'arrêt du Conseil d'État cité par les auteurs de l'amendement, il est justement précisé que le préfet ne peut pas être « moins disant » que la loi sur ce point, en ayant une interprétation restrictive de l'extension.

C'est la raison pour laquelle un équilibre doit être préservé entre la réponse à des besoins légitimes en logement et la sauvegarde des activités agricoles. La présente proposition de loi conditionnait initialement l'autorisation de nouvelles constructions dans les zones en principe inconstructibles à leur compatibilité avec des activités agricoles et forestières. Le présent amendement vise à réintégrer ce garde-fou. ? Les assouplissements que le texte propose d'apporter visent principalement la construction dans les hameaux, autour des corps de ferme et en bordure de village. Par essence, ce sont aujourd'hui des terrains « gelés », car ils sont classés comme espaces agricoles au sein de ces communes rurales, même lorsqu'ils ne sont pas directement exploités.

est classée en zone agricole. Je crains que cette condition supplémentaire n'interdise, par exemple, à un exploitant agricole de se loger sur son exploitation, ce qui aurait pour conséquence de restreindre trop fortement la portée de l'assouplissement proposé dans le texte. En outre, les parcelles incultes ou sous-exploitées ne sont pas identifiées d'un point de vue urbanistique ; il sera donc difficile de les caractériser dans un PLU.

n'est pas définitif. D'autre part, il a pour objectif de permettre à un tiers de demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale,

n° 18 rectifié. Cet amendement vise à permettre au règlement du PLU des communes concernées de fixer des règles de base applicables aux constructions proposées.

dans le règlement du PLU la mention précise des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, à condition toutefois de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère. Cela n'a rien à voir ! L'application de cette disposition

Même avis, monsieur le président.

amendement vise à renvoyer au décret le soin de fixer un cadre commun pour déterminer les « communes peu denses en déprise démographique » et dont le territoire fait l'objet de fortes contraintes urbanistiques, c'est-à-dire celles qui bénéficieront des assouplissements prévus par le présent article. Comme nous l'avons décidé en commission, ce sont les intercommunalités qui affineront le ciblage, mais il faut une base de travail commune et objectivable.

l'objectif de « développement économique et démographique de l'ensemble du territoire, dans les communes urbaines comme rurales ». En m'inspirant des avancées obtenues par le Sénat dans le cadre de la loi Climat et résilience, je propose de garantir que les objectifs chiffrés des SCoT en matière de lutte contre l'artificialisation et de consommation d'espace prendront en

je l'ai souligné en commission, je pense que le « Denormandie dans l'ancien » est un excellent outil, qu'il nous faut prolonger au-delà de sa période initiale de trois ans, jusqu'en 2025. Pour autant, avant d'envisager une prolongation de près de trente de trente ans, il nous faut d'abord conduire une évaluation en bonne et due forme, avec l'appui de la Cour des comptes, et examiner les résultats du dispositif sur les dix premières années, par exemple. C'est un principe de responsabilité et d'évaluation des politiques publiques, que nous devons à nos concitoyens. Par ailleurs, si nous voulons donner une vraie impulsion et lancer une dynamique forte pour la réhabilitation du bâti ancien en zone rurale, mieux vaut prévoir une date butoir proche, plus incitative qu'une échéance très lointaine. Pour ces raisons, la commission demande le retrait

plutôt qu'à la construction, alors que nous disposons d'un vivier important de bâtiments vacants. L'article 4 prévoit d'en limiter l'extension aux communes peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance. Or ces biens rénovés seront destinés non pas à l'acquisition, mais à la location, ce qui pourrait être inadapté pour ces territoires. Il serait plus pertinent de créer un dispositif fiscal spécifique

les zones connaissant un fort taux de vacance. Il écarte donc les communes rurales peu denses, qui ne disposent pas d'un tel parc de bâtiments disponibles. Afin de ne pas pénaliser ces dernières, le présent amendement vise à supprimer le critère relatif au fort taux de vacance pour bénéficier de l'extension du Denormandie dans l'ancien.

c'est-à-dire celles qui bénéficieront de l'extension du Denormandie dans l'ancien. Les intercommunalités affineront ensuite le ciblage, comme pour le « Pinel breton

comment caractériser concrètement les besoins en logement ? En outre, l'adoption de cet amendement aurait pour effet de centrer les aides fiscales sur les zones tendues, soit exactement l'inverse de ce que nous souhaitons. Il faut encourager la modernisation de l'habitat dans les zones rurales. Cet amendement tend aussi à supprimer le mécanisme de territorialisation, inséré en commission, par lequel les intercommunalités d'un département contribuent à identifier les communes rurales qui bénéficieront de la mesure.

de la dégradation du bâti en zone rurale. Je ne souhaite pas supprimer ce critère utile au ciblage de la mesure. Par ailleurs, la territorialisation du dispositif inséré en commission permettra de cibler plus finement les communes éligibles, par exemple en vérifiant les raisons de la vacance.

Le développement du logement social agricole nous semble ainsi très intéressant. Des initiatives se développent pour que des bailleurs sociaux achètent des maisons d'habitation liées aux exploitations agricoles, les rénovent le cas échéant et les louent ensuite aux agriculteurs. Toutefois,

Un rapport du Gouvernement sur ces initiatives permettrait d'identifier les pratiques présentes sur le terrain et les politiques publiques efficaces pour les soutenir. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement,

commission ? L'adoption de cet amendement étendrait significativement la portée de l'article 5, aujourd'hui strictement limité au logement nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation. Seraient ainsi autorisées toutes les activités artisanales connexes,

et dès lors qu'elles « ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ». L'activité fromagère que vous citez en défense de votre amendement répond à ces critères.

ou à proximité de celle-ci, quel que soit le classement du terrain d'emprise au regard du document d'urbanisme applicable. Les auteurs de la proposition de loi présentent cette mesure comme « le droit pour chaque agriculteur à vivre sur son exploitation Toutefois, il nous semble que cette mesure risque encore une fois de créer de l'habitat diffus. Le terme « à proximité » étant relativement flou, nous proposons de le remplacer par « en continuité », en cohérence avec les dispositions du code de l'urbanisme sur ces questions.

qui restreignent encore davantage les espaces cultivés en zone périurbaine. Cette pression engendre de nombreux conflits d'usage entre agriculteurs et nouveaux riverains. La création des zones de transition entre espaces artificialisés

Une fois de plus, champs, vignes et vergers battent en retraite face aux lotisseurs. Vous en conviendrez avec moi, ce débat a un caractère quelque peu schizophrénique : d'un côté, nous voulons préserver nos exploitations agricoles et notre indépendance alimentaire ; de l'autre, nous voulons à tout prix urbaniser des zones pour favoriser l'habitat rural sur des terres agricoles

de situations particulières, après avis favorable de la CDPENAF.

on fait tout l'inverse ! Je m'étonne que, pour régler des conflits de voisinage ou d'usage, on retire ainsi des terres agricoles à l'agriculture. Les agriculteurs sont d'ores

C'est un vrai sujet, j'attire votre attention

Le scrutin est ouvert.

En effet, tous les sénateurs ruraux le constatent régulièrement, des nuisances ou des troubles de voisinage reconnus par la loi sont utilisés à l'encontre d'exploitations agricoles. Certes, la loi et la jurisprudence reconnaissent ce droit, puisque le code civil

du droit de propriété, une théorie spécifique au cas particulier des troubles anormaux de voisinage. Ainsi, sous certaines conditions, le juge judiciaire accepte d'indemniser les nuisances considérées comme excédant les inconvénients normaux du voisinage. Sur le fondement de ce principe, on peut donc solliciter réparation, que l'on soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Contrairement à la responsabilité du fait personnel, le recours en indemnisation sur le fondement de troubles anormaux de voisinage n'exige pas la démonstration d'une faute quelconque.

M. Daniel Salmon. Si nous sommes sensibles à la question soulevée par cet article- la protection des agriculteurs face à de potentiels recours abusifs du voisinage contre leur exploitation nous estimons que la rédaction retenue et les conditions dans lesquelles est discutée cette disposition ne permettent pas de prendre une décision adéquate. C'est pourquoi nous proposons sa suppression. En effet, l'article exclut les troubles liés à une activité agricole préexistante du champ des dommages ouvrant droit à réparation dans le cadre d'un recours des voisins. Sa rédaction est proche du droit existant, mais ne précise pas que les activités agricoles doivent s'exercer dans le respect de la réglementation en vigueur, ce qui semble plus que problématique. En outre, si des recours abusifs ont pu être constatés sur ce sujet, le droit existant reste protecteur, la reconnaissance de la pré-occupation. Comme l'a souligné la commission des affaires économiques, il convient d'être très vigilant à la réforme de cette disposition, dans la mesure où toute exonération de responsabilité en matière de troubles de voisinage touche à des principes constitutionnels forts. telle vigilance a également été rappelée par le Conseil d'État, qui estime que l'état actuel du droit permet d'ores et déjà d'assurer une protection équilibrée des intérêts en présence et qu'il ne paraît pas nécessaire de modifier profondément les équilibres existants.

l'exigence de poursuite des activités agricoles « dans les mêmes conditions » est assouplie, afin de permettre une évolution à la marge des pratiques agricoles liées, par exemple, à l'évolution des machines agricoles ou à la variation des cultures.

Il s'agit de prévenir d'éventuels recours abusifs de la part de nouveaux arrivants à l'encontre d'agriculteurs préalablement installés et exerçant leur métier dans le respect de la réglementation. L'article 113-8 du code de la construction et de l'habitation répond, dans une certaine mesure, à l'objectif visé par cet article, tout en précisant que les activités concernées doivent se poursuivre dans les mêmes conditions. Si une telle précision peut se comprendre pour les autres activités visées, industrielles, commerciales ou touristiques, elle se justifie moins pour les activités agricoles qui évoluent sensiblement dans le temps. Le présent amendement vise donc à modifier le droit en vigueur en créant une distinction entre les activités agricoles et les autres.

d'une intervention trop tardive de ces commissions, d'un manque de lisibilité de leurs critères d'examen, voire d'une forte variabilité de leurs avis entre territoires ou entre dossiers. Tout cela contribue à dégrader l'acceptabilité de leurs décisions. Pourtant, elles jouent un rôle crucial pour la préservation des terres agricoles et des forêts françaises.

et les définitions qu'elles retiennent. Ensuite, un rapport du Gouvernement analysera l'ensemble de ces lignes directrices pour évaluer si des mises en cohérence sont nécessaires et si de bonnes pratiques peuvent être partagées. Certaines CDPENAF ont déjà amorcé ce travail. Cet amendement vise à le généraliser et à l'approfondir,

observations ? ... Il en est ainsi décidé. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à définir